Cette ouverte. Le compte rendu analytique de président séance a été distribué. Je ne vois pas d'observation et donc adopté sous les réserves d'usage. Je veux dire collègues et je dois vous informer qu'que le président du Sénat n'a été saisi d'aucune opposition à la demande de création d'une commission spéciale sur la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification, l'extension du risque incendie. Dans le délai prévu par l'article 16 du règlement conséquence c'est ce bis par mois. En conséquence cette proposition de loi est renvoyé pour son examen à une commission spéciale. Lors du jour appelle maintenant. Les réponses à des questions orales. La parole est à monsieur Alain Milon. Pour sa question.-- Merci monsieur le président. Madame la ministre, la loi 2021 1017 relative à la à la bioéthique du 2 août 2021 a ouvert l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes célibataires et à instituer. La possibilité de congés leurs gamètes sans motif médical ce droit très attendue s'avère difficile à mettre en oeuvre en effet le code de santé publique réserve ce droit de procéder aux prélèvements on recueille à la conservation des gamètes au 16 établissements publics de santé et aux établissements de santé privés à but non lucratif Or l'ouverture des techniques d'AMP à toutes les femmes génère une forte augmentation de l'activité médicale et c'est tant mieux, elle accroît le nombre de demandes de sperme et une pénurie de don de gamètes et redouté principalement causée par la levée partielle de l'anonymat des donneurs de ce fait, les centres d'AMP risquerait de ne plus être en mesure de satisfaire l'ensemble des demandes et d'ores et déjà le délai d'attente. De prise en charge des patientes ont largement augmenté, faute de moyens supplémentaires cette certes l'article L 21 41 tiré 12 du code de santé publique prévoit que par dérogation si aucun organisme ou établissements de santé publics ou privés à but non lucratif n'assure ses activités dans un département, le directeur de l'ARS peut autoriser un établissement privé. À but lucratif de les pratiquer, sous certaines conditions. Cela ne répond nullement aux besoins liés à l'afflux de demandes. J'aimerais donc Madame la Ministre savoir s'il existe une possibilité d'élargir en supprimant les conditions dérogatoires aux établissements de santé privés à but lucratif. Le droit de pratiquer ce prélèvement le recueil la conservation diamètre on l'pesant évidemment les mêmes contraintes et obligations qu'aux autres établissements.-- Merci cher collègue. Madame le Ministre. Merci monsieur le président. Mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Alain Milon. Le Ministre de la Santé François Braun regrette de ne pouvoir être présent ce matin et et m'a demandé de vous fournir. Les éléments de réponse suivants. Alors vous l'avez dit, hein, cette loi du 2 août 21 relative à la bioéthique étant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées et c'est une avancée sociétale majeure. Le nombre de demandes émanant de couples de femmes et de femmes non mariées se situe à un niveau très supérieur à ce qui avait été anticipé. Aux propos sur le 1er trimestre 22, plus de 9000 demandes ont été enregistrées. Alors que l'hypothèse la plus haute envisagée dans l'étude d'impact, s'établissait à 4000. Donc le stock de gamètes, fait l'objet d'enquêtes régulières de l'Agence de biomédecine. Tout comme le niveau d'activité, les délais de prise en charge et les moyens engagés, il n'y a à ce jour aucune pénurie de spermatozoïdes, a déploré le nombre de donneurs continuent de s'accroître. À la faveur notamment de campagnes de sensibilisation. Le gouvernement a, par, par ailleurs mis en place un financement exceptionnel en aide à la contractualisation non reconductible de 7 millions, 3 en 2021, à destination des centres pour leur permettre de faire face à l'afflux de de monde cet accompagnement financier s'est poursuivie en 2022 et il se pérennise en 2023 par un financement lui pérennes donc. Sous forme d'une mission d'intérêt général AMP. Ces mesures ont permis de limiter la hausse des délais d'accès qui sont passées de 13 mois huit à 12 mois en décembre 21. Et j'ajoute que le gouvernement lance actuellement des concertations pour optimiser l'offre à législation constante et réduire les délais d'attente. Concernant le, la place du secteur privé lucratif. Je veux quand même rappeler que la structuration du secteur est fondée sur le régime de la gratuité et du volontariat du don. Seuls les établissements publics ou privés non lucratifs peuvent être autorisés pour le don de gamètes ou d'embryons et il en est de même pour l'activité d'auto-conservation sans motif médical peut-on faire évoluer cela il faudra conserver le régime de la gratuité et du volontariat. C'est bien là la question. Voilà. Madame la ministre. Monsieur Milan. Merci. La parole est à présent monsieur Philippe mouiller.-- Merci monsieur le président, madame le ministre, ma question porte sur les conséquences de l'application du décret numéro 2022, de 157 du 22 février 2022 pour les personnes en situation de handicap qui occupent un emploi. En effet les dispositions de ce décret relatif au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d'invalidité ont des conséquences particulièrement injuste pour les travailleurs handicapés. Depuis l'apparition de ma question orale au Journal officiel du Sénat. Je suis assailli de témoignages de personnes dont la situation personnelle est directement impacté par ce texte. Que prévoit ce décret. Il a introduit une nouvelle méthode de calcul des pensions d'invalidité. Le plafonnement au plafond annuel de la Sécurité sociale passe du salaire de comparaison. Par conséquent les personnes invalides, dont les revenus d'activité dépassent le Pass. Voit le montant de leur pension d'invalidité suspendu. Ce qui entraîne de facto et c'est peut-être là le plus important, la suspension des rentes de prévoyance puisque ces dernières sont assujetties au versement d'une pension d'invalidité alors que certains ont cotisé depuis de nombreuses années. Les travailleurs en situation de handicap. Titulaires d'une pension d'invalidité ont vu leur versement de celle-ci, suspendu. Depuis la parution de ce décret et donc depuis le mois de septembre 2022 et ce, sans avoir été informée en amont. En raison de la perte totale des versants de leur pension. Certaines d'entre elles ne se dans une situation financière délicate. D'autres envisagent même de cesser toute activité professionnelle alors que le travail est synonyme dispensé passion et d'indépendance financière. Ce texte réglementaire va manifestement à l'encontre de l'esprit de la réforme qui vise à favoriser le cumul emploi-ressources et globalement des politiques d'emploi pour les personnes handicapées aussi je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer les mesures que vous entendez prendre afin de remédier corriger améliorer ce qui est vécu pour les intéressés comme une véritable discrimination. Je vous remercie.

effectivement. En avant le fait d'avoir, de favoriser la reprise d'activité, vous l'avez dit. Auparavant, la pension d'invalidité qui compenser la perte de gain ou de capacité de travail. Étaient calculés sur les revenus moyens des 10 dernières Années civile de salaire actuellement c'est calculé en fonction de ce salaire de comparaison de ce seuil, de la sécurité de plafond de sécurité sociale qui est 3666 euros brut par mois en 2022. Ce salaire de comparaison est un choix de cohérence qui tient au fait que la pension d'invalidité est une prestation sociale. Et que toutes les prestations sociales sont prises en compte à partir de revenus plafonnés. Par ailleurs, la réforme n'entraîne plus une réduction systématique et parfois total du montant de ce dépassement avec le seuil de comparaison puisqu'elle permet aujourd'hui ce cumul partiel entre revenus d'activité et pension d'invalidité alors aujourd'hui 60.000 pensionnés d'invalidité. Ont vu leurs revenus s'améliorer avec ce décret du mois de février. Mais il y a effectivement des personnes c'est toujours le cas dans ce type de de mesures à peu près 7000, soit un peu moins de 3% des invalides du régime général qui exercent une activité professionnelle, qui ont vu une réduction de leur pension. Donc le service du ministère de la Santé de la prévention étudie actuellement ces situations particulières. Qui nous sont remontés afin que nous puissions trouver les meilleures. Les meilleures solutions pour elle. Mais sur un plan général, le régime adopté et tout de même favorable à la majorité des personnes pensionnés. Merci la ministre maintenant, la parole est à monsieur Guy Bénard Roche. Merci monsieur le président, ma question s'adresser au Garde des Sceaux, ministre de la justice et concerne la généralisation des cours criminelles départementales, les délais d'audiencement soit beaucoup plus court en matière de violences sexuelles et sexistes. Nous avons mis à terme aux insupportable correctionnalisation telle était la réponse du milices le 13 décembre lors d'une question de ma collègue écologiste à l'Assemblée vous interrogeant sur la généralisation des CCD vous connaissiez Monsieur le Ministre de position au sujet des jurés populaires. Il sort plus qu'important car il concrétise le principe d'être jugé par ses pairs. Selon une loi pénale votée par ses représentants. La position de refus d'une généralisation du l'expérimentation d'en évaluer que nous avons pu exposer accompagner nos craie d'une justice spécialisées dans les violences sexistes et sexuelles qui ne dirai son nom ni ne bénéficierait d'une réelle spécialisation et formation la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a fait un pas en prévoyant la généralisation. En place à comité d'évaluation des CCD dont j'ai été moi pour le Sénat. Les résultats ne sont pas ceux qui ont été avancés. Rien ne vous permet de conclure que cela a mis un terme aux corrections égalisation que de regrettant tout autant que vous le directeur des services judiciaires a lui va Madické de pas être en mesure d'établir le nombre de dossiers concernés et leader des syndicats des magistrats indique que aucune baisse de la charge des audiences correctionnelles a été constatée. Le rapport conclut que le comité partage le constat général d'une difficulté d'évaluation de l'impact des CCD sur la correctionnalisation et souhaite qu'une étude soit menée à sept fait et propose de doter la DACG d'un outil statistique lui permettant d'appréhender les effets du fonctionnement de ces CD sur la correctionnalisation. Ma question porte plus particulièrement sur point d'attention constant que j'ai pu porter haut c'est des travaux de ce comité. Les besoins en ressources humaines inhérents à la généralisation. Le comité a mis en évidence les Il a par ailleurs à Londres de retour d'expérimentation qui ne fait état que de 9% des affaires qui se déroule devant cinq magistrats de carrière souhaitait qu'une évaluation du nombre de magistrats et de greffiers rendue nécessaire au fonctionnement généralisé des CCD dans les conditions prévues par la loi, soit. Avant la mise en oeuvre de cette généralisation, la généralisation est officiellement en place depuis le 1er janvier. Pouvez-vous donc Monsieur le Ministre, nous donner cette évaluation demander des besoins RH, ces chiffres mettent fois réclamé.-- Madame la Ministre.-- Merci monsieur le président, monsieur le vice-président de la commission des lois. Monsieur le garde des Sceaux me me me charge de de répondre à cette question. Et le gouvernement et comme vous particulièrement attaché aux jurés populaires. C'est pourquoi la souveraineté du jury populaire dans les cours d'assises a été renforcée par la loi confiance en décembre 2021, puisqu'il faut désormais une véritable majorité de jurés pour condamner un accusé. Le rapport du comité d'évaluation dont vous faites partie a été rendu en octobre 22 et permet de conclure que les objectifs poursuivis par cette expérimentation liés notamment à la réduction des délais de traitement de procédure qui criminels sont globalement atteint l'ensemble des personnes y compris les plus critiques à la vue à l'égard des cours criminelles départementales s'est accordé pour reconnaître que les principes de l'oralité des débats et du contradictoire avait été respectées comme en cour d'assises les plots les plaidoiries se déroule dans un climat moins pesant. Les parties civiles étaient plus à l'aise pour s'exprimer dans cette nouvelle juridiction. Et les délais d'audiencement sont plus courts 12 mois contre 18 mois pour une cour d'assises. La CDD cour criminelle départementale permet en effet de juger les crimes dans des délais beaucoup plus rapides que les cours d'assises et permet de restituer aux faits de viol massivement correctionnel lisez leurs véritables qualification les CDD juge 81 pour 81% des affaires de viol concernant les besoins de magistrats du à cette généralisation, j'indique que les magistrats honoraires et magistrats à titre temporaire ont pleinement joué leur rôle. 74% des affaires jugées. Le collège des magistrats était composé de deux magistrats honoraires et à titre temporaire, soit le nombre maximum permis par la loi, ainsi dans ces cas les affaires mobilisé 3 magistrats soit autant qu'une audience correctionnelle par, par ailleurs, ces magistrats sont professionnels et sont renforcés par les avocats honoraire ayant des fonctions juridictionnelles créé par la loi confiance et qui peuvent composer ce collège de magistrats en CCD ce nouveau statut a rencontré un franc succès chez les avocats, le garde des Sceaux travaille bien sûr avec les professionnels du droit et les universités pour intensifier tous ces recrutements. Beaucoup Madame la Ministre Monsieur Mison hein maintenant la parole.-- Merci, monsieur le Président Madame le Ministre initialement. Ma question s'adressait à Monsieur le Ministre de la Santé. La commune de folle comment en Moselle est prête à lancer un projet innovant et atypique qui consiste à développer un village de l'autonomie et du handicap dans son centre-ville concrètement des logements adaptés, sécurisés permettrait aux résidents de ce village de bénéficier des services de la ville dans les 2 domicile de continuer à profiter pleinement d'une vie sociale grâce à la proximité de commerce ou encore de participer à diverses activités l'ensemble comprendrait 24 pavillon senior de Pavio de colocation pour 16 résidents. Une structure de réadaptation pour personnes âgées vieillissantes qui pourrait accueillir 30 personnes hébergement permanent et temporaire confondus et enfin une maison d'accueil médicalisé de 33 places, le tout entraînerait la création de 70 emplois-qui favoriserait la la revitalisation de ce bourg chef-lieu de canton en milieu rural, pour les 30 prochaines années. Or bien que tout soit réglé au plan financier des difficultés administratives freinent sa réalisation. L'ARS ne délivrant pas les autorisations nécessaires aussi et vous en avez le pouvoir. Je vous le demande solennellement, madame la ministre, pouvez-vous débloquer ce dossier et le faire enfin aboutir. Et. Merci cher collègue. Madame la Ministre, vous avez la parole pour 2 minutes je rappelle. monsieur le président, Monsieur le Sénateur. Mison. Avant de répondre sur cette situation particulière que vous évoquez, je je tiens à rappeler et vous le savez que les autorisations délivrées par les autorités de contrôle et de tarification le sont uniquement lorsque les projets sont de qualités qui correspondent aux orientations du projet régional de santé et qu'ils répondent à un besoin étayé et prioriser sur le territoire concerné, ce sont les seuls critères qui guide les éventuelles décisions. Je souligne également que toute ARS et par principe, à l'écoute des projets émergents sur les territoires et les accompagne au regard de ces règles. Le projet de village, de l'autonomie et du handicap de folle mon est un projet composite. Vous l'avez dit, hein. Dont certains éléments d'ailleurs ne relève pas des compétences de l'ARS. 2 aspects le concerne néanmoins un aspect avec une maison d'accueil médicalisé de 33 place par la Fondation personnage il y a eu une rencontre organisée par l'ARS, avec la fondation personnelle je le 17 mars 2022, en présence du maire de la commune et du conseil départemental de la Moselle. Il a été indiqué par l'ARS de Moselle que. À l'heure actuelle à ce jour là il n'y avait pas de possibilités de financement parce que les agréments entraîne forcément des financements des autorités vous le savez, qu'il n'y avait pas à ce jour de de possibilités de financement et que ceux-ci ne pouvait être attribué que par appel à projets après examen de toutes les candidatures, ne sait pas, ne s'est pas manifesté à nouveau auprès de l'ARS. Mais malgré ces informations partagées, il semble que des engagements était anticipée peut être par des élus du territoire en dépit de ses réponses. Une autre partie du projet concerne la construction d'une structure de réadaptation pour personnes handicapées vieillissantes, porté par une association gestionnaire. Qui sollicitent une participation ARS. Là aussi, une réunion a eu lieu en juillet 22 une nouvelle réunion aura lieu le 2 février 23. Afin de faire avancer ce projet. je veux rappeler très simplement que ces projets doivent correspondre donc à un besoin territoriale partagé entre le conseil départemental l'ARS et les organisations gestionnaires, qu'il faut avoir bien sûr les crédits disponibles et qu'il faut répondre à des appels d'offres qui sont lancés par l'ARS et le conseil départemental et c'est dans ces conditions que les projets pourront voir le jour et être agréé. Un mécanisme monsieur en. Merci monsieur le président me la ministre, nous n'avons pas le même niveau d'information. Moi je sais que cette commune travaille depuis 4 ans sur ce projet et qu'à l'heure où on. On essaie d'accélérer les procédures dans certains secteurs, je trouve que. Dans ce domaine. Le, l'administration a quelque peu à la du retard. Moi je pense que l'administration est là pour répondre aux attentes de rendre service aux porteurs de projets

Lance son appel à projets et la commune. Il répondra. Très rapidement.-- La parole était présent au président Pierre Laurent.-- Merci monsieur le président, madame la mini-j'attire aujourd'hui votre attention sur la situation de l'hôpital de La Roche-Guyon dans le Val-d Oise. Établissements spécialisés dans l'accueil du polyhandicap pédiatrique. Nous attirons régulièrement j'étais a alerté par cette sur cette situation par des syndicalistes à l'Automne lors de ma visite à l'hôpital Trousseau dont dépend la Roche-Guyon. Nous attirons régulièrement ici la tension avec les professionnels sur la situation de de l'hôpital singulièrement dans la dernière période sur la situation. Des services de pédiatrie. Mais là nous sommes sur le cas spécifique de l'hôpital de La Roche-Guyon. Un hôpital dans lequel la multidisciplinarité des professionnels médicaux et paramédicaux en font un lieu de vie quotidien et d'hospitalisations unique pour des enfants. À la hauteur des besoins de soins nécessaires pour des enfants. Polyhandicapés, or l'hôpital connaît des difficultés structurelles de recrutement, de formation, de conditions de travail et de salaires trop bas qui conduisent à la fermeture permanente de lits dans cet hôpital et la difficulté de recrutement et renforcé à La Roche-Guyon par la situation géographique de l'établissement son isolement en matière de transports publics et son et le déficit de logements sociaux abordables à proximité pour le personnel. Malgré les efforts de la direction et de l'encadrement médical et paramédical. Environ 10 lits sur 80 sont fermés depuis plus d'un an et d'autres sont menacées, si la situation perdure et c'est pour ces raisons je vous serais reconnaissant de m'indiquer ce que l'État. En coordination avec tous les acteurs concernés entend entreprendre en vue de remédier à cette situation extrêmement périlleux préjudiciable pour un établissement dont la fonction est unique. Merci. Merci beaucoup madame la Ministre.-- Merci monsieur le président. Monsieur le vice-président. Oui, le l'hôpital de La Roche Guyon connaît des difficultés de recrutement. Malheureusement comme beaucoup d'établissements sanitaires. De notre pays à l'heure actuelle et ses difficultés de recrutement, on tenait impact sur l'activité et ont effectivement conduit à fermer une dizaine de lits temporairement. Il s'agit pour l'essentiel, de difficultés d'attractivité des métiers que nous connaissons France entière et non de fidélisation. La quasi-totalité des agents de l'hôpital habite à proximité de l'hôpital avec un coût de l'immobilier qui est quand même bien inférieur à celui par exemple de Paris intra-muros. Si l'établissement rencontrent des difficultés à recruter. Il convient toutefois de noter que les agents, une fois qu'ils sont recrutés reste assez durablement en poste dans ces établissements et que tous les agents bon n'utilise pas de transport en commun parce qu'il n'existe pas. Certainement mais viennent travailler en voiture et que la question des transports publics. N'est pas ce qui ressort le plus dans leurs besoins. Un plan de réouverture progressive des lits a été engagé devant permettre d'ouvrir la totalité des 80 lits de la structure d'ici l'automne 2023 au fur et à mesure des recrutements d'infirmiers. Pour ce faire différentes mesures d'attractivité sont engagés par l'établissement. L'hôpital propose des contrats d'allocation d'études pour les infirmiers, infirmières ou mais par exemple à disposition des logements. Ça a été le cas pour des masseurs kinésithérapeutes. Ce qui a contribué au recrutement de 4 kiné ces derniers mois alors qu'il n'y en avait plus aucun à l'été 2022. Je souligne également l'ouverture d'une nouvelle unité. Au mois de novembre 22 qui consiste en une extension de l'hôpital dans un bâtiment neuf et cette nouvelle unité permet d'offrir aussi aux patients des meilleures conditions de prise en charge et au personnel des meilleure qualité de vie au travail qui renforce ainsi l'attractivité de l'hôpital et sa capacité à fidéliser. Donc ce sont des mesures locales auxquelles viennent s'ajouter bien sûr des mesures plus larges portés depuis 4 ans par l'ARS Île-de-France sur les ressources humaines en santé sur ce territoire francilien. 50 millions d'investissements en faveur du logement des soignants 400 contrats allocation études par an ou encore un million cinq pour financer des formations d'IDE qui. Devenir. IPA donc des infirmiers en pratique avancée, donc oui nous devons continuer à travailler sur l'attractivité de ces métiers. Si beaucoup madame la Ministre, Oui. Très rapidement, je vous invite. Toutefois, à ne pas minimiser la situation. C'est du temporaire. Vous l'avez dit mais du temporaire qui dure et qui dure depuis trop longtemps, alors que les besoins sont considérables. Donc vous pouvez compter sur moi, sur les syndicalistes qui sont d'ailleurs présents aujourd'hui. Pour rester vigilant sur cette situation et. Suivre l'évolution promise. Par vos. Votre réponse ce matin. Merci madame la ministre. les conditions d'éligibilité aux paiements Directs découplé ont été détaillées par le ministère par les services du ministère de l'agriculture. Sur cette base à travers vous, madame, j'appelle l'attention Monsieur le Ministre de l'Agriculture. C'est la mauvaise prise en compte des surfaces collectif d'alpage dans l'application du plan stratégique national la nouvelle politique agricole commune effectif donc au 1er janvier de cette année en l'état actuel des critères retenus par l'éco-régime, seul le gestionnaire pourrait directement touchés l'liée à l'éco-régime sur les surfaces de la page collectif. Ceci est contraire au mode de calcul des aides découplées pour lesquels des portions de surface collectifs sont réaffectés à chaque éleveur en fonction du nombre d'animaux conduits sur la dite de surface au prorata du temps passé sur l'espace collectif. Une telle situation conduit à des pertes d'aides importante pour les éleveurs et va mettre à mal leur trésorerie tout en provoquant une inégalité de traitement entre les alpages privé les alpages collectif dans la démarche écologique et pourtant plus marquée par ailleurs une grande partie des alpages collectif de mon département, les Hautes-Alpes sont gérées par des syndicats. Or le plan stratégique national ne les reconnaît pas juridiquement comme gestionnaire éligible aux aides européennes de du premier pilier. Vous connaissez l'importance Madame la Ministre des pratiques pastorales dans mon département et plus globalement de l'élevage. Dans ces conditions, quelles sont les mesures correctives qui peuvent être envisagées par le gouvernement et le ministère de l'agriculture pour faire face à cette problématique. contribuera je n'en doute pas à soutenir les éleveurs. Je vous demande donc d'être à côté de nos éleveurs et nos agriculteurs je vous remercie. Merci, monsieur le Président. Je vous prie d'excuser Monsieur le Ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, qui m'a demandé. De vous répondre et je le fais avec un grand plaisir. Monsieur le sénateur vous attirer notre attention sur ce plan stratégique national. aux dispositions applicables aux surfaces pastorales qui ont été et au coefficient d'admissibilité de ces surfaces et très technique mais c'est important pour les agriculteurs qui ont été maintenus à un niveau inchangé. L'éco-régime doit permettre de valoriser les services environnementaux rendus par l'élevage extensif. C'est pourquoi il a été décidé de l'étendre aux mécanismes de rapatriement des surfaces d'estive gérés en commun par les éleveurs bénéficiaires de cette aide au prorata de leur utilisation en cours d'année. Ce mécanisme avait déjà été mobilisés dans le cadre du versement de l'aide de base pour un développement durable. Le respect des critères conditionnent le versement de l'éco-régime sera vérifié d'une part sur les surfaces déclarées par l'exploitant dans son dossier PAC conformément à la voie d'accès choisie par le demandeur et d'autre part sur les surfaces rapatrié d'estive, conformément à la voie d'accès s'appliquant à ces surfaces utilisées en commun le gestionnaire d'estive pourra selon le même principe, faire une demande d'aide et obtenir le versement de l'éco-régime. Il faut souligner que du point de vue réglementaire, un agriculteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personne physique ou morale ayant une exploitation et exerçant une activité agricole donc un syndicat gestionnaire d'estives peut donc répondre à cette définition. S'agissant du caractère actif le PSN et le décret du 31 décembre 22 relatives aux aides de la PAC définit l'agriculteur actif selon que le demandeur d'aide est une personne physique une société une structure de droit public ou encore une association pour ce qui concerne les gestionnaires d'actifs leur éligibilité à ce caractère d'agriculteurs actifs s'appréciera donc à la lumière de la forme juridique de la structure porteuse du collectif. pour les syndicats intercommunaux dont on sait qu'ils peuvent être gestionnaire d'estive, ce sont les établissements publics de coopération intercommunale. C'est donc une forme de personne morale de droit public, il est bien prévu par le PSN dans les formes répondant à la définition d'agriculteurs actifs c'est très technique mais je crois que ça répond à la majorité des cas. Merci monsieur Arnaud.-- Oui madame Annie, je vous remercie. D'après les premiers éléments que vous des nos connaissances doivent satisfaire l'ensemble des acteurs de la filière et et des estives de mon département et au-delà de tous les départements français et je tenais à vous en remercier.

La mise en oeuvre de cette réglementation présente de réelles difficultés. En l'absence d'outils efficaces de suivi de l'utilisation des sols. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'articuler cette réglementation avec d'autres, comme celles relatives aux plantations de sapins de Noël aux règles strictes de hauteur d'âge ou encore de densité pouvant conduire à passer d'une qualification du culture à une qualification de boisement cette situation s'observe ainsi dans le département de la Nièvre 1er producteur de sapins de Noël. Le département en l'absence d'outils facilement mobilisables se retrouve vite démuni dans l'exercice de cette mission de suivi de l'utilisation des sols. Or pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune. L'État s'appuie sur le registre parcellaire. Graphique Neaud N. Non anonymisé mise à jour aujourd'hui tous les 3 ans, a suivi satellitaire devrait permettre à l'avenir une actualisation annuelle découvert. Aussi pourrait-on mettre à la disposition des départements les informations non-anonymisé relatives à ce registre parcellaire graphique, s'il n'est pas peu si se dégrade pas possible madame la Ministre, pourriez-vous me dire dans quelle mesure l'État pourrait traiter ces informations pour le compte des départements. Je vous remercie. Collègue Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le le sénateur joli. Alors les cultures de sapin de Noël en pleine terre ne sont pas admissibles aux aides de la politique la politique agricole commune. Vous, vous l'avez dit jusqu'en 2022 inclus le régime le registre parcellaire graphique le fameux RPG ne permettait pas de les identifier. Il est prévu que les exploitants puisse les déclarer en 2023 comme culture non admissibles. Toutefois, cette information ne sera en aucun cas exhaustive, elle sera limitée aux seuls déclarant Pâques qui auront souhaité détailler des cultures non admissibles dans leur déclaration. La localisation des parcelles concernées sera ensuite publié chaque année par l'IGN sous la forme d'une cartographie nationale détaillé et anonymisé. Le RPG contenant des données personnelles et relevant du secret des affaires sa réutilisation est soumise au droit relatif à la protection des données personnelles, ainsi qu'aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que ces informations ne sont pas communicables Ne sont de miser pardon ne peut par conséquent pas être mis à la disposition des départements. Néanmoins, dans le cadre de ses missions de service public et en cas de nécessité avérée les conseils départementaux peuvent se rapprocher des directions générale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt pour convenir des modalités de traitement de ces données par leur service afin de répondre au mieux à leurs besoins.-- Oui, monsieur le président, mes chers collègues. Madame la ministre. Ma question porte sur la crise pédiatriques dans le Cher. Une question que j'espérais vous présenter plus tôt. Et en effet, comme de nombreux territoires non notamment ruraux le Cher souffrent de d'une pénurie de pédiatres. Et pour vous exposer la situation à ce jour, le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges. Ne dispose que de 3 praticiens. Dont un qui s'approche de la retraite et un autre qui est à 80%. La situation est telle que la seule unité de néonatologie. Théologie avec soin intensif du département installé à Bourges risque de fermer. Alors je sais que vous allez me dire il y a un plan d'urgence de 150 millions d'euros. Bon et assez. J'en doute, d'autant que nous ne savons toujours pas comment cette somme sera déployé. De surcroît, c'est une action très coûte court-termiste et je ne suis pas sûr que ce soit des millions d'euros qu'il faut mais aujourd'hui ce sont des pédiatres. Aussi je souhaite savoir comment allez vous agir pour endiguer cette urgence dans mon département, lequel est déjà fortement touchée par le problème plus général de la désertification médicale. Mais là il s'agit de l'accès aux soins pour nos enfants, petits-enfants nos nourrissons. Nous sommes dans une impasse ou leur santé et mise en jeu. Merci monsieur le président, Monsieur le le sénateur pointe euros bon vous me faites par des difficultés rencontrées en pédiatrie dans le département du Cher et et vous l'avez dit, c'est le cas dans de très nombreux départements ruraux en particulier dans notre pays. Et bien sûr nous devons apporter des réponses à court terme et puis aussi envisager le moyen terme et le long terme. Alors à court terme, le centre hospitalier de bourgeons sait qui connaît une situation de tension sur ses effectifs de pédiatres, du fait notamment d'arrêt de maladie de maternité, entre autres, cette situation est connue de l'Agence Régionale de Santé qui est très mobilisé pour soutenir les professionnels et garantir la plus haute qualité de soins. Les équipes du centre hospitalier ont su trouver des solutions pour assurer la permanence des soins notamment au cours des week-ends d'octobre dernier, où les plannings n'étaient plus remplies et où la situation a pu apparaître la plus difficile. Je souhaite profiter de cette réponse pour saluer la mobilisation de la communauté hospitalière pour répondre aux besoins de leurs patients à fortiori lorsqu'il s'agit de prendre en charge des nourrissons et des très jeunes enfants. Une partie de la réponse a pu être retrouvée grâce à une collaboration avec la clinique Guillaume II varie de Bourges où les praticiens qui exercent. tout le monde a été. Mis en responsabilité sous l'égide de l'ARS et ses efforts témoigne de la mise en place une coopération intelligente entre les structures publiques et privées qui là encore réfléchissent collectivement pour assurer une prise en charge efficace des patients sur le territoire. Alors ça, bien sûr, monsieur le sénateur, vous l'avez dit, c'est dur, court terme. Il faut que ce soit du court terme le plus court possible au moyen terme. Vous le savez un pédiatre il faut le former le numerus clausus a été levée et il nous faut des années de formation, donc nous devons pendant ce temps là, être. Le plus pertinent possible et surtout. Trouver des des solutions les plus. Les plus structurés les plus pertinentes pour les territoires avec tous tous les professionnels de santé du territoire, ce qui a été fait à Bourges et qui continuera d'être fait. Merci, madame la Ministre, Monsieur, mon cher collègue.-- Oui Madame la Ministre j'entends bien ce que vous dites mais c'est vrai qu'il nous faut des solutions. Concrètes et et de de court terme, parce que la coopération avec Guillaume de varices et c'est vraiment au cas par cas. Et et de court terme, il faut qu'on ne nous formions davantage de pédiatres le numerus clausus a peut-être augmenté mais on n'a pas augmenté. La filière de de pédiatres. Donc c'est vrai que le cher et est un département où la désertification médicale et et toujours s'enracine dans le dans on alerte en permanence le le gouvernement sur ce sujet mais moi je prie pour qu'il n'y ait pas j'ai pas vous interpeller un jour madame la mise sur la la suite à la suite d'un drame quoi c'est ce que je vous, je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. Merci cher collègue. Maintenant, la parole est à madame Dumas.-- Merci monsieur le président, ma question s'adresse aux monsieur, à monsieur le ministre de l'Intérieur. Madame la ministre, en concertation avec le maire du XVIIe arrondissement de Paris. Geoffroy Boulard je souhaite aujourd'hui attirer votre attention sur le niveau insuffisant des effectifs du commissariat du 17e arrondissement situé rue lors du précédent quinquennat, le président de la République avait fait de l'augmentation des effectifs des forces de sécurité, une priorité. Avec le projet de recruter près de 10.000 fonctionnaires supplémentaires. Cette mesure allait de bon sens au regard de la multiplicité des missions affecté à la police nationale. Après 5 ans de mandat Ford, force est de constater que cette promesse ne s'est pas traduite concrètement dans les fêtes, notamment dans notre arrondissement. En effet, malgré la création, l'année dernière d'une brigade équipés de vélo terrain on constate depuis plusieurs mois une baisse constante des effectifs jusqu'à atteindre un niveau critique l'été dernier où pendant toute la période estivale. Le XVIIe n'a disposé en soirée que d'un seul véhicule police secours ainsi depuis 2017 les effectifs ont diminué de 15%. Et bien que la préfecture de police dispose de plusieurs unités qui peuvent venir en soutien de notre commissariat lors d'opérations de police spécifique. Ces unités ne sont pas présentes au quotidien dans l'arrondissement pour concourir à la sécurité des habitants. Or le 17ème arrondissement compte près de 167.000 habitants, il doit faire face à un important problème de sécurité dans un bon nombre de quartiers. Il relève donc de la responsabilité de Monsieur le Ministre de l'Intérieur de fournir les effectifs suffisants pour permettre aux fonctionnaires de la police nationale de réaliser au mieux leur mission et ainsi protéger nos concitoyens. Nouveau préfet de police de la capitale. Laurent Nunez nous a annoncé l'affectation de 1000 nouveaux policiers. L'installation de 500 nouvelles caméras alors Madame la Ministre qu'en est-il de ces informations, pouvez-vous nous rassurer sur ce point, les élus et les habitants demandent arrondissement l'attendent avec impatience.

de 283 fonctionnaires parmi lesquels 252 membres du corps d'encadrement et d'application plus six policiers adjoint le modèle d'organisation de la préfecture de police présente la particularité d'intégrer sous l'autorité du préfet de police. L'ensemble des services de police oeuvrant à la sécurité des Parisiens. Ce modèle spécifique a une conséquence directe. Il est impossible de se limiter au seul effective d'un commissariat d'arrondissement pour mesurer les moyens mobilisés pour assurer les missions de sécurité publique. La direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne la DSP AP a en charge les commissariats parisiens leurs effectifs sont variables suivant les arrondissements en fonction de la population et des enjeux de sécurité propre à chacun, mais la DS P gère aussi des sous-directions spécialisées qui contribuent directement à la sécurité des habitants du XVIIe arrondissement, la sous-, direction de la police des transports qui oeuvrent dans le métro et le RER, la sous-, direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, la sous-, direction des services spécialisés qui abrite en son sein des compagnies de sécurisation et d'intervention et les brigades anti-criminalité. D'autres directions spécialisée de la préfecture de police peuvent agir au sein du XVIIe arrondissement pour gérer les problématiques particulières toujours en lien avec le commissariat local. La direction de la police judiciaire avec ces brigades centrales sa sous-, direction des affaires économiques et financières et ses divisions territoriales est notamment chargé des investigations judiciaires sur le spectre haut et moyens de la délinquance de la criminalité organisée et du terrorisme. Donc la la direction de la police judiciaire. Je viens de citer. La direction de l'Ordre public maintenant et et de la circulation, spécialisée dans la protection des institutions, la sécurité, la circulation routière et le maintien de l'ordre public, c'est-à-dire l'encadrement de toutes les manifestations de voie publique à Paris. Troisièmement, la direction du renseignement qui assure la fonction de renseignement territorial et participe à l'action de prévention et de lutte contre le terrorisme avec en particulier le suivi des individus radicalisés et puis pour finir, la direction de l'innovation de la logistique et des technologies qui apporte un support logistique à l'ensemble des directions de la préfecture de police. Les directions de police administrative contribue également à la préservation de la sécurité de minutes et de la tranquillité publique, ce sont bien toutes ces directions au-delà du pivot du pivot que constitue le commissariat d'arrondissement qui concourt à la mise en rayon des actions en faveur de la sécurité des Parisiens, pardon monsieur le président. Mais mais largement dépassé. Je pense qu'il est indispensable que vos collaborateurs prépare des réponses. Qui correspondent au délai qui est prévu par le règlement du Sénat. Monsieur Lenglart. Vous avez la parole.-- Merci, monsieur le Président. Madame la Ministre le 10 janvier 2022. Le président de la République a annoncé la création de 200 brigades de gendarmerie en milieu rural. Cette annonce a trouvé une suite dans le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur voté définitivement au Sénat au mois de décembre 2022. L'augmentation du budget de la sécurité intérieure va permettre la création de postes supplémentaires et la création de nouvelles brigades la densification du maillage territorial de la gendarmerie et nécessaire dans l'objectif de rapprocher les forces de l'ordre de la population que les nouvelles brigades soit fixe ou qu'elle prenne la forme d'unités itinérantes. Les Brigades fixe seront adossés soit la mise à disposition de bâtiments existants, soit à la réalisation de projets. Ces nouvelles brigades de gendarmerie devront être opérationnel d'ici 5 ans. Ce ce délai interpelle d'un temps la mise en oeuvre ce projet soulève des difficultés ce délai interroge au regard des difficultés que je constate en Aveyron. En effet l'annonce de la construction d'une caserne de gendarmerie AS pas Lyon date du 23 septembre 2020, soit 2 ans avant l'annonce du président de la République et la loi Lopmi. Elle devrait être envisageable, à court terme, mais encore faudrait-il que ce projet avance, et avance vite. Ce qui n'est pas le cas depuis 2 ans cette caserne et qui est nécessaire pour España, Lyon et le nord Aveyron va offrir des conditions de travail plus satisfaisante aux militaires et de meilleure qualité de vie à leurs familles ce qui favorisera également de l'économie locale. C'est pourquoi madame la ministre, je vous interroge sur 2 points. D'une part, pouvez-vous apporter des précisions concernant les rénovations et constructions prévues en Aveyron, dans le cas de la création de 200 brigades de gendarmerie en milieu rural et d'autre part quelles sont les informations concrètes sur l'avancée de la gendarmerie de Lyon. Que les élus et les gendarmes attendent depuis longtemps. Quand est-ce que les gendarmes pourront l'occuper je vous remercie. la sécurité des Français en garantissant une plus grande proximité une présence de voie publique accrue et une meilleure prise en charge des victimes. Les préfets en lien avec les commandants de groupement de gendarmerie départemental conduisent actuellement une large concertation avec les élus dans les territoires pour déterminer les modalités de création de ces unités en tenant compte des enjeux identifiés dans chaque département, cette phase de concertation lancée en septembre 2022 se déroulera jusqu'en février mars 2023, elle permettra d'examiner les propositions faites par les élus, en prenant en considération à la fois les besoins opérationnels de la gendarmerie nationale, l'offre immobilière disponible les conditions de travail et de vie. Ainsi que la mobilisation locale autour du projet. Les propositions formulées aboutiront après analyse par les échelons locaux et centraux aux premières décisions au cours du 1er trimestre 2023 s'agissant de la construction de votre caserne. J'ai envie de dire d'une caserne de gendarmerie sur la commune d'Espagne on et sur le fondement d'un agrément de principe immobilier délivré en octobre 2020 mais services ont agréé en novembre 2022 le futur terrain d'assiette et les conditions juridiques de l'opération issus des dispositions du décret du 26 décembre 2016. Il appartient désormais au maître d'ouvrage désigné en l'espèce l'entreprise sociale pour l'habitat sud Massif Central habitat de produire les compléments d'information financiers juridiques attendu et de s'engager résolument dans la phase de conception technico-architectural du projet sur la base des référentiels qui lui ont été communiquées sur cette base l'autorisation de lancement des travaux devraient permettre une livraison de la nouvelle caserne fin 2025. Si le chantier se déroule de façon nominale, partie prenante dans ce montage la mairie d'espalier on est et restera et je. M'engage à éveiller systématiquement informé des échanges entre le, la gendarmerie de l'Aveyron et le maître et le maître d'ouvrage afin que tous les partenaires de cette opération immobilière et connaissance de l'état d'avancement du projet. Voici monsieur le sénateur, les éléments que je souhaitais vous avoir. Madame la Ministre. C'est OK pour le collègue maintenant, la parole est aux questions, Jean-Pierre Sueur.-- Merci, monsieur le Président Madame la Ministre je voulais appeler votre attention sur le statut des correspondants de presse. En effet, comme vous le savez depuis la loi du 27 janvier 1987. Qui leur a conféré la qualité de travailleur indépendant. Aucune évolution de leur statut n'a eu lieu. Cette loi. Dispose notamment que le correspondant local de presse je cite contribue à la collecte de toute information. qui dans les faits et celui des correspondants de presse alors que leur rémunération et la prise en charge leurs frais sont très limitées. J'ajoute qu'il n'y a pas de grilles tarifaire que les correspondants locaux de presse ne cotisent pas à l'Urssaf et qu'ils ont donc un statut très précaire, alors qu'il participe pleinement à la rédaction à la mise en forme et à la diffusion de l'information auprès de nos concitoyens, en outre, dans nombre de publications. Il ne dispose pas de la possibilité de signer leurs articles, ce qui a pour effet d'anonymiser un travail intellectuel, personnel. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous demander ce que le gouvernement compte faire. Afin de faire évoluer le statut des correspondants de presse pour qu'ils correspondent mieux à leur activité réelle.

ma collègue de la Culture m'a chargé de vous répondre. La presse régionale et départementale joue un rôle déterminant pour la vitalité de la vie démocratique local l'activité des correspondants locaux de presse, vous l'avez souligné, est à ce titre totalement central pour que l'actualité soit couverte au plus près des territoires en application des dispositifs. De l'article 10 de la loi numéro 87 39 du 27 janvier 1987, modifié par l'article 16 de la loi 93 121 du 27 janvier 1993. Les correspondants locaux de presse sont des collaborateurs occasionnels des titres de presse locale. Leur activité leur permet en principe et pour la majorité d'entre eux de percevoir des revenus à titre accessoire en complément d'une autre rémunération comme par exemple une pension de retraite. Les correspondants locaux de presse non pas. Donc vocation à se substituer aux journalistes professionnels salariés par les titres auxquels ils contribuent ou à se voir appliquer des dispositions applicables aux journalistes professionnels. La loi du 27 janvier 1987 leur a conféré le statut de travailleur indépendant qui leur permet d'imputer sur leur bénéfice imposable les charges professionnelles nécessaires au fonctionnement de leur activité tels que par exemple les frais de déplacements et ces professionnels bénéficient également d'un régime dérogatoire de cotisations sociales, soutenue par le budget de l'État. Je vous précise en conclusion que pendant la crise sanitaire, l'État et les régions mis en place différents dispositifs d'aide aux travailleurs indépendants dont les conseillers locaux de de presse afin d'amortir une baisse de leurs revenus. Je vous remercie.-- je. Connaît ses correspondants de presse puisque je les rencontre. Tout le temps sur le terrain dans les déplacements dans les communes et je peux vous dire qu'ils assument un travail important qu'ils remplissent des pages de nos. Journaux Journaux régionaux. Avec une rémunération tant de leurs déplacements que de leurs articles et leurs photos qui est extrêmement faible, donc je réitère. Auprès de vous et de Madame la Ministre de la Culture et de la communication. Leur souhait de voir leur statut amélioré.-- Merci. Là maintenant à madame Florence l'actrice. Monsieur le Président Madame la Ministre le spectre des coupures électriques semble s'éloigner. Pour l'instant, grâce aux efforts de sobriété, de nos concitoyens mais aussi grâce aux températures anormalement élevées de cet hiver qui témoignent malheureusement du changement climatique. demeure fragile avec de nombreuses centrales de production électrique à l'arrêt pour une longue période, les risques de délestages pour cet hiver ou l'hiver suivant ne sont donc pas. Aussi les élus locaux que nous sommes pour la plupart d'entre nous demeure-t-il très vigilant et inquiet. Nos associations notamment l'Association des maires de France, la Fnccr vous ont alerté depuis des mois sur la situation des stations d'assainissement et de traitement d'eau potable. Des coupures d'électricité sur ces sites pourraient avoir des conséquences majeures pour les habitants. Coupures d'eau dans les hôpitaux bornes d'incendie inutilisables pollution dans les milieux naturels en effet concernant l'eau potable, même si les réservoirs sont le plus souvent recharger la nuit, des coupures d'électricité ferait peser des risques notamment sur les installations de reclodée, passion au fil des réservoirs néanmoins indispensable pour assurer la potabilité de l'eau. Concernant l'assainissement, les risques de pollution en cas de coupures d'électricité sont bien réelles dans les stations de traitement mais aussi dans les postes de refoulement, avec des risques de déversement d'eaux usées non traitées dans les milieux naturels, avec des délais de prévenance court il est par ailleurs difficile d'imaginer des groupes électrogènes spécifique et indépendant pour chacune de ces installations aussi, j'insiste à nouveau pour que ces installations indispensable soit classé en installation prioritaire dans le cas contraire, comment l'État par l'intermédiaire de ses services déconcentrés accompagne-t-il les collectivités responsables de l'eau potable et de l'assainissement dans la préparation de céder les stages et enfin, quel sera le régime de responsabilité en cas de pollution liée au délestage. Les élus sont inquiets à Madame la Ministre. Merci cher collègue. Madame la ministre à vous.-- Merci monsieur le le président, madame la sénatrice bla triste compta. Comme vous le savez notre notre pays traverse sa plus grande grave crise énergétique depuis les les chocs pétroliers des années 1970. Nous avons pris depuis l'été et continuons de prendre toutes les dispositions nécessaires pour passer l'hiver dans les meilleures conditions possibles. Cela passe notamment par la maximisation des moyens de production. La sécurisation de nos importations et notamment l'accès l'accélération des projets d'énergies renouvelables et la reconduction de notre consommation d'électricité. Nous souhaitons d'ailleurs remercié les Français pour leur mobilisation sur le mois de décembre, la baisse de consommation retraités les températures étaient de 8 5 %, c'est considérable. Cette mobilisation a porté ses fruits et notre système électrique a pu surmonter la vague de froid de décembre tout en maintenant un signal EcoWatt verts. Même si nous abordons l'hiver dans les meilleures conditions, notamment. Avec les 13 réacteurs arrêtés le 6 janvier soit une disponibilité supérieur au scénario central de RTE et des températures pour le moment 12 l'hiver n'est pas terminée et nous devons continuer à nous préparer à des scénarios extrêmes dans lesquelles du délestage pour être nécessaire. La réglementation prévoit que les installations prioritaires sont inscrites dans la limite d'un plafond de consommation totale au niveau départemental sur des listes afin de ne pas être coupé la priorité absolue étant d'éviter les menaces immédiates sur la vie d'une personne. Les installations d'eau potable et d'assainissement ne sont pas explicitement prévu par l'arrêté du 5 juillet 1990 encadrant ces listes d'usagers dits prioritaires. Pour autant, cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas prises en compte dans l'exercice de priorisation. À l'échelon local réalisé par les préfets. La situation dépend de chaque territoire. Le gouvernement et les préfets ont conduit un travail avec plusieurs filières et les gestionnaires du réseau électrique afin d'examiner les situations particulières notamment la filière de l'eau et de la scène l'assainissement pour leur permettent de se préparer au mieux au risque de coupures en l'occurrence ici pour identifier leurs sites les plus à risque et y concentrer leurs moyens de sécurisation. Nous pouvons passer un hiver sans coupure. Ce sujet est l'affaire de tous, opérateurs, État, collectivités territoriales, élus, acteurs économiques et associatifs et citoyens eux-mêmes je vous remercie.

Madame la secrétaire d'État. La pêche guyanaise se meurt. Elle se meurt, qui plus est sous nos yeux. Faute de rentabilité. Sur les 130 laissant de licences de pêche côtière. Seuls 45 100 régulièrement exploitées. Pourtant la Guyane fait sans doute partie des derniers espaces maritimes les plus riches en ressources halieutiques de l'Europe bleue. Les mots sont connus vétusté de la flotte, absence de oeuvre pêche illégale. Des solutions existent, mais les bonnes décisions ne sont pas prises ou le son avec retard alors qu'il y a urgence d'agir. Madame la secrétaire d'État. Où en sommes-nous des études sur la ressource un préalable. Ben pourtant imposé par l'Europe au renouvellement de la flotte. On en parle depuis 2017. L'urgence c'est la pêche côtière, celle qui nourrit les Guyanais et qui fait tourner les usines de transformation. À quand les premières constructions et avec quel type de bateau. Quid du plan d'action de 2018 qui proposait également la création d'une nouvelle flotte pour exploiter la bande des 30 à 200.000 nautiques inexploité aujourd'hui quelle est la réponse à notre demande d'aller vite en récupérant les navires sorti de la faute de pêche de La Manche suite au Brexit dans une démarche d'économie circulaire où est le blocage. Concernant le nous rouge seul secteur à résister qui a perdu la franchise de taxes douanières de 15% suite à une réécriture malheureuse d'un règlement européen les démarches auprès de la commission ont-elles été initié la problématique de la concurrence déloyale, organisé par l'Europe avec les périphériques pêcheries des pays ACP a-t-elle été déposée. Enfin concernant la pêche illégale, il faut une surveillance, 7 jours sur 7, tous les bateaux quittant les eaux guyanaises devrait contrôler et les mesures de saisie, destruction des navires de pêche illégale systématiser. Il en va de la survie du secteur et c'est aussi une question de souveraineté de l'État. Madame la secrétaire d'État, les enjeux liés à la pêche sont importants, vitaux pour le territoire. La Guyane dispose d'un potentiel. Dans le passé. Dans les années 90 à 2000 avec 140 navires pour la pêche côtière et 83 chalutiers pour la pêche au large. Nous avions déjà une pêche compétitive. Le port du pêche du Larivot, chers collègues. Était alors de. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre mettons en place et vite les moyens.-- Madame la ministre, qui se souvient que le délai de réponse et de deux minutes.-- Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les les sénateurs, monsieur le sénateur patients. Déjà, je vous prie d'excuser l'absence du secrétaire d'État chargée de la mer. Hervé Berville qui n'a pas pu être présents ce matin. Nous connaissions monsieur le le sénateur les difficultés subies par les pêcheurs guyanais et par évidemment la la pêche illégale, notamment. C'est un phénomène structurel de grande ampleur est un véritable fléau pour la Guyane et plus largement pour la France si nous sommes le 2ème espace maritime mondial. C'est d'abord et avant tout grâce à ses outre-mer et le gouvernement ne peut donc pas se satisfaire des difficultés que connaissent les territoires comme vous, le gouvernement veut une filière locale de pêche qui soit rémunératrices durable et un levier pour le développement économique de votre territoire et pour l'activité des populations locales. C'est pour cette raison que mon collègue Hervé Berville a demandé au directeur général des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture, de se rendre en Guyane en décembre afin de lancer un cycle d'échange sur ces sujets avec tous les acteurs du secteur maritime guyanais. L'État déploient déjà des moyens considérables dans la lutte contre la pêche illégale 300 contrôles par an réalisé par la Marine nationale, la gendarmerie et les Affaires maritimes. L'État va encore augmenter ses efforts à la suite de ce déplacement, le secrétaire d'État a d'ores et déjà lancé 2 actions concrètes sur la pêche illégale la première la construction d'une nouvelle unité côtière pour les Affaires maritimes la deuxième la signature d'une convention avec le comité régional des pêches de Guyane Liffey maire est également WWF pour la réalisation d'une étude sur l'impact économique de la pêche illégale. Concernant les droits de douane sur le vivaneau rouge le règlement européen sur les contingents tarifaires autonome pour certains produits de la pêche sera prochainement renégocier l'évolution de son contenu devra se faire en cohérence avec les intérêts des autres régions ultra-maritimes qui ont développé une production locale de vivaneau.--

Merci monsieur le président, madame la ministre, ma question s'adresse au ministre des Transports. Mais vous êtes là donc. Merci de les prendre à ma question qui concerne le prix exorbitant des billets d'avions d'avions pardon, qui ne cesse d'augmenter pour les territoires d'outre-mer la hausse observée sur les 12 derniers mois et de l'homme du recours, les voyageurs au départ et à destination de nos territoires doivent débourser plus de 30% de plus qu'il y a un an, ce qui impacte considérablement le budget des ménages qui souhaitent se déplacer pour des raisons familiales, économiques ou professionnelles. Cette réalité du prix excessif des rotations aériennes depuis ou vers les Outre-mer n'est pas nouvelle et l'asphyxie nos populations et s'amplifie d'année en année et s'inscrit dans un phénomène structurel de Vie chère en Outre-mer et de situation monopolistique déjà ancien, aux racines historiques et aux conséquences humaines dramatiques cette conséquence cette conséquence est irréversible, quelques fois pour les familles qui ont des moyens limités, est devenue insupportable et intenable. Donc aujourd'hui nous souhaitons et je demande que qu'il y ait un bouclier tarifaire sur les prix. Concernant la continuité territoriale aérienne pour les outre-mer à l'instar de ce qui se fait déjà en Corse. Il conviendrait également de mettre en place une politique ambitieuse d'ouverture du ciel en décentralisant les autorisations d'ouvertures de lignes aériennes souvent bloqués par la direction générale de l'aviation civile. L'objectif est de faciliter la concurrence qui allie, ce qui ça en tout cas au renforcement des instances de contrôle introduit par la loi du 20 novembre 2012 relatives à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer permettant de jouer poser positivement sur la concurrence, mais aussi la formation des prix et qu'on viendrait également et surtout de plafond mener les prix pour les outre-mer pour les billets pour que ce ne soit pas au-delà de 500 euros, aujourd'hui on a des billets dans la classe économique qui sont à plus de 1000 euros ça va donc Merci madame la ministre, c'est à vous.-- Tout d'abord les routes aériennes entre la métropole et les départements d'outre-mer sont des liaisons européennes et à ce titre, entièrement libéralisés donc toute compagnie française ou européenne peut librement les exploiter. Les prix des billets d'avion vers les départements d'outre-mer ont augmenté de 8% entre 2019 et 2022, légèrement moins que l'évolution constatée au départ de la métropole, sur l'international long-courriers qui elle est près de 12%. Cette hausse est notamment due à la hausse du prix des carburants plus 94% entre les mois de septembre 2021 et septembre 2022 et des augmentations plus fortes localement comme aux Antilles. Qui n'a pas été donc intégralement reportés sur le prix des billets et de manière générale à l'inflation. Les liaisons vers les départements outre-mer sont néanmoins plus concurrentiel que l'ensemble des autres liaisons long- courrier, notamment du fait de la présence d'un nombre important de transporteurs 3 compagnies exploitent les vols vers les Antilles et quatre vers la Réunion.-- Enfin, nous souhaitons rappeler l'action de l'État en faveur de la continuité territoriale, le fond de continuité territoriale finance notamment le passeport mobilité études le passeport mobilité en stage professionnel le passeport mobilité formation professionnelle et l'aide à la continuité territoriale. Au total, l'État a consacré près de 16 millions d'euros à ces dispositifs. En 2021, le choix a été fait de soutenir de manière renforcée les personnes fragilisées par l'augmentation des prix et pour cela, la loi de finances pour l'année 2023 renforce les moyens de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité ce qui limitera le reste à charge des bénéficiaires des aides à la continuité territoriale à 50% du prix du billet. Les collectivités qui ont la compétence sociale peuvent aussi fixer les tarifs sociaux. Merci chéri, madame la Ministre, pardon. Et maintenant, la parole est à Édouard Courtial. Madame la Ministre. Personne ne conteste que la lutte conte l'artificialisation des sols soit désormais bien identifié comme un enjeu prioritaire pour la préservation de l'environnement et la biodiversité. Personne non plus ne serait prêt à revenir sur l'objectif zéro artificialisation nette d'ici 2050 et la réduction de moitié en disons qui ont été inscrits dans la loi climat et résilience. Si le fond n'est donc pas un sujet il y a en revanche beaucoup à redire sur la forme. Malgré les nombreuses mises en garde du Sénat, notamment lors de l'examen du texte brutal centralisatrice. Irrespectueuse des différences territoriales irréaliste punitives. Les mots des élus locaux ne sont pas assez dur pour définir la méthode employée. Comment le leur reprocher lorsqu'aucune ingénierie aurait proposé pour les accompagner et qu'ils se sentent une fois de plus abandonnés par l'État. Comment le leur reprocher lorsqu'ils constatent une fois encore, une façon de faire descendante depuis Paris qui refuse le bon sens du terrain. Comment le leur reprocher. Lorsque les décrets sont plus restrictif que la loi entretenons un flou juridique à leur désavantage. Pourtant nous avons dans cet hémicycle voter une Terrier réalisation de l'objectif et nous avons demandé de faire confiance aux élus tout simplement un revirement a enfin été amorcée par le gouvernement 7h car nécessaire compte tenu des enjeux et de l'inquiétude des élus. Ainsi Madame le Ministre, êtes-vous favorable au prix utilisation du Sénat notamment celle exprimée dans une PPL transpartisane déposé le 14 décembre dernier, qui se décline en 3 axes assouplir le calendrier des documents d'urbanisme ne pas obérer la capacité foncière des collectivités initions des grands projets structurants et enfin instaurer une territorialisation Dusan pour aider les petites communes rurales. Je vous remercie. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les les sénateurs, monsieur le sénateur Courtial. Vous avez interrogé monsieur Christophe Béchu Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, ne pouvant être présent il m'a chargé de vous répondre. Chaque année, 20.000 hectares d'espaces agricoles naturels et forestiers sont consommés en moyenne en France, soit près de 5 terrains de football par heure. Tous les territoires sont concernés, y compris les territoires ruraux. Sur la dernière décennie, la consommation d'espace et d'ailleurs majoritairement localisés sur les territoires détendu, plus particulièrement en péri-peu dense à très peu dense. L'esprit de la réforme et de diminuer pour l'avenir la consommation nationale des espaces naturels et agricoles tout en continuant à assurer un développement des territoires qui en ont besoin pour cela, la France s'est fixé l'objectif d'atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050 avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers dans les 10 prochaines années. Cette trajectoire progressive, elle a décliné dans tous les documents de planification et d'urbanisme la territorialisation de la trajectoire dans les, dans ces documents devra moduler le rythme d'artifice. D'artificialisation des sols en tenant compte des besoins et des enjeux locaux dynamique démographique économique équilibré du territoire. Cette dernière dimension comprend les enjeux de désenclavement rural. Le 24 novembre dernier, la Première ministre a réaffirmé qu'il fallait garantir que toutes les communes rurales puissent bénéficier d'une possibilité de construction en particulier lorsqu'elles ont peu construit par le passé. Prévoir un décompte des projets d'envergure nationale à l'échelle nationale encore. Ces différents ajustements devraient trouver une déclinaison en 2023 dans le cadre de travaux menés avec les parlementaires et les représentants des collectivités territoriales pour accompagner les collectivités. Le gouvernement a aussi renforcer l'offre en ingénierie locale en étendant les missions des établissements publics fonciers des agences d'urbanisme et de la haine. C'était en faveur de la sobriété foncière. Je vous remercie.--

pour saluer le volontarisme affiché et exprimer à l'instant, pas Madame le Ministre mais lui redire aussi la vigilance qui sera la mienne pour que ça Stasiulis concrètement sur le terrain. Merci monsieur le président. Monsieur maintenant a vraiment la parole La crédibilité de la parole de l'état du gouvernement et donc je vais respecter la chronologie. Le 14 octobre 2021. Le maire de la commune de Lambersart m'a alerté sur la difficulté rencontrée dans le cadre du dispositif alvéoles les 5 abris à vélos commandé en mai 21 ne pouvaient être livrées par la société. Abris plus dans le délai imparti par le dispositif de subventions. Ce retard était dû selon le fabricant à la pénurie de matières premières à la forte demande de tels équipements et puis aussi on était en période de de Covid le 20 octobre 21, j'ai envoyé un courrier à Madame Pompili, ministre de la transition écologique afin de lui demander l'obtention d'un sursis auprès du dispositif alvéoles la ville Lambersart ayant rempli son dossier dans les temps impartis. Le 30 novembre 2021 en séance publique au Sénat. Madame bah secrétaire d'État chargée de la biodiversité m'assurer que les dossiers non complet à cause de la pénurie de matériel seraient étudiée en priorité et avec bienveillance, dans le cadre de alvéoles plus ça valait engagement le 1er septembre dernier, j'étais à nouveau interpellé par monsieur Bush, maire de Lambersart l'AFUB lui a annoncé que ces dossiers ne figurait pas sur la liste d'attente des bénéficiaires éligibles à la au projet alvéoles Monsieur le maire a relancé l'AFUB afin d'avoir plus d'explications à ce sujet, mais à ce jour, aucune réponse ne lui a été fait. Alors je réitère ma demande car le dispositif est intéressant et toutes les communes devraient pouvoir en profiter, surtout si elles ont effectué les démarches dans les délais impartis. Est-il possible que le gouvernement intervienne comme le ministre s'y était engagé comme la ministre qui était engagé en faveur d'un assouplissement du dispositif alvéoles plus au profit de la commune de Lambersart mais aussi de beaucoup d'autres donc au bénéfice du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique. Je vous remercie, madame la Ministre.-- Merci Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les les sénateurs, monsieur le le sénateur. Le programme alvéoles visait à aider les collectivités locales à installer des stationnements vélo sécurisés en s'appuyant sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Ce programme a été un succès à la fin du programme. Décembre 2021, près de 18.000 emplacements sécurisés ont été installés. Grâce à son soutien dans un contexte d'augmentation de l'usage du vélo par les Français à la fin de la crise sanitaire, les demandes d'aide se sont concentrés au cours des derniers mois d'éligibilité. Engageant la fin de ce programme. Le ministère de la transition écologique a retenu un nouveau programme c'est. Sur le même thème. Au cours de l'année 2021 avec un volume augmenter pour viser 100.000 emplacements. Les porteurs du programme ont organisé la gestion de la forte demande des 6 derniers mois d'alvéoles pour le dans l'objectif de satisfaire le plus de bénéficiaires possible. Cela a été menée dans un contexte de périodes de fin de pandémie sanitaire mais aussi de tensions internationales sur les approvisionnements des matières premières. Les services du ministère de la transition écologique ont demandé que les porteurs informe régulièrement les bénéficiaires de l'état de leur demande d'aide et évalue les difficultés rencontrées lors de la réalisation de leurs projets. Cette communication a été menée au plus tôt en 2021, et de manière régulière avec les bénéficiaires 322 demandeurs ont ainsi été suivis individuellement afin de mener à leur terme les projets malgré des demandes tardives et des retards de délais d'approvisionnement de leur projet. Suite aux échanges avec les porteurs. 289 ont reçu une réponse favorable dans le cadre du programme alvéoles plus qui prolonge les actions relatives au stationnement vélo ce qui représente donc 90%. La commune de Lambersart à solliciter une demande d'aide pour l'installation de 3 stationnement sécurisés de vélo en date du 5 juillet 2021, période de fin de programme dès le dépôt de la demande d'aide. La commune a été informé que celle-ci s'inscrivait dans une liste d'attente au vu de la forte demande et que le versement de l'aide n'était pas assuré. La commune Lambersart s'inscrivait dans la liste des dossiers des 322 demandeurs les porteurs du programme en sollicité à plusieurs reprises la commune pour connaître l'état d'avancement du projet. Celle-ci n'a pas répondu aux sollicitations des porteurs et n'a pu bénéficier des aides. Je suis trop courte. Je vous donnerai les, les détails de la fin de la réponse. Monsieur le sénateur. Si beaucoup Madame la Ministre.-- La parole maintenant est à monsieur Gillet. remercie monsieur le Président Madame la Ministre. La modification du périmètre de site Natura 2002 Garonne en Nouvelle Aquitaine et source d'incertitude pour les agriculteurs et populi culteurs concernés en vallée de Garonne cette extension répondant aux enjeux définis dans la stratégie nationale de biodiversité l'inclusion au sein d'un site Natura 2000 ne signifie pas l'adhésion car les démarches d'engagement existantes sont basés sur le volontariat. Lorsqu'un signataire s'engage, il doit mettre en oeuvre des pratiques cohérente envers les orientations du document d'objectifs favorable à la biodiversité par ce biais peut bénéficier de certains avantages financiers. La principale interrogation de ces acteurs agricoles et populiste. Réside dans l'éventuel durcissement de la réglementation en vigueur, notamment relatives aux couples de peuples. Et au 1er boisement peupliers en site Natura 2000, régi par les listes locales, départementales. Par ailleurs, ils sont également concernés par la réglementation relative aux retournements de prairie rejet également par les listes locales, départementales, ainsi que pour les cultures par le projet de décret relatif à l'encadrement sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en site Natura 2000 terrestre suite à la décision du Conseil d'État du 15 novembre 2021. Il nous semble pas opportun de mettre en place des restrictions complémentaires alors que des outils contractuels existent déjà, comme les contrats agricoles et Charte pouvant être engagée comme sur la Garonne depuis plusieurs années. Ces restrictions complémentaire risquerait d'être contre-productive vis-à-vis de l'animation territoriale des gens en place depuis depuis ces années. Pouvez-vous nous confirmer que les prochaines évolutions réglementaires. S'il y en a prendront en compte ces enjeux économiques en accompagnant ses agriculteurs et populi culteurs dans leur pratique et ne créeront pas de contraintes réglementaires supplémentaires sur le site Natura 2000, je vous remercie. Merci monsieur le le président, mesdames, et messieurs les les sénateurs, monsieur le le sénateur gilet. La France s'engage fortement en faveur de la protection de la biodiversité, notamment au travers des objectifs fixés par le président de la République dans la stratégie nationale pour les aires protégées. Nous souhaitons couvrir le territoire national par un réseau cohérent d'aires protégées à hauteur de 30% du territoire. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement ne fait pas contre, mais avec les partenaires sociaux économiques. Ainsi le modèle français de Natura 2000 n'exclut pas a priori les activités économiques présentes dans les sites. Le régime d'évaluation des incidences est fondé sur un système de liste au niveau national et départemental, l'extension du site Natura 2000 peut en effet aboutir à soumettre certaines activités qu'n'y était pas soumis jusque-là à une évaluation des incidences cependant l'existence des listes départementales de projets et activités soumis à évolution des incidences Natura 2000 est due à la volonté de prendre en compte les enjeux locaux sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 et d'éviter que des formalités administratifs ne soit requise inutilement la même logique de subsidiarité a présidé à la rédaction du décret relatif à l'encadrement de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000, les préfets étant compétent pour les encadrer leur utilisation lorsque cet encadrement n'a pas été prévu par les chartes et contraint. La France pour la gestion des sites Natura 2000 à privilégier la contractualisation. Les propriétaires des terrains inclus dans le site peuvent conclure des contrats comportant un ensemble d'engagements conforme aux orientations définies par le document d'objectifs, sur la conservation ou le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du du site restant fidèle au mode contractuel que la France a choisi pour mettre en oeuvre la politique Natura 2000, l'accompagnement des acteurs reste la voie privilégiée.-- Si Madame la Ministre le sénateur Gilles dispose d'un crédit. Gens. Je vous remercie, merci pour votre réponse. Madame la Ministre vous l'avez compris. Il y a des inquiétudes, mais en même temps une volonté d'engagement donc il faut accompagner effectivement les les parties prenantes. Et peut être travailler sur les temporalités pour rassurer. Et faire en sorte que ces engagements puisse se mettre en place dans les meilleures conditions possibles mais il faut prendre en considération cette inquiétude qui est effectivement légitime. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Laurent Bureau Merci, monsieur le Président Madame la Ministre l'Observatoire du Mont-Aigoual fait partie des plus anciennes stations de France et du monde. Néanmoins, devant les avancées technologiques. Cette dernière fermera au 31 mars 2023. Mais au printemps 2023 s'ouvrira un centre d'interprétation et de sensibilisation au changement climatique, géré par la communauté de commune Causses Aigoual Cévennes terre à solidaire ce futur centre s'appuie sur une Exposition permanente et dès 2005. Ce projet a su convaincre et c'est avec le soutien des collectivités du département de la région et même de l'État que des travaux conséquents de réhabilitation ont été engagées en 2019 et pour un montant de 3,5 millions d'euros. Aussi, la communauté de communes a souhaité élargir son soutien au delà de la saison estivale en proposant des activités éducatives et en accueillant des séminaires ce Champ d'action prend en compte l'activité Centre de tests en conditions climatiques extrêmes que météo France ne souhaite plus poursuivre et qui s'adresse à des essais. L'entreprise industrielle aux chercheurs et j'en viens alors ce qui m'interpelle dès sa conception, le projet s'est constitué autour de la mise à disposition de personnel espère de météo France pour assurer la médiation scientifique principe AT par l'ancien PDG de météo France à 2019. Cet engagement s'est traduit dans le projet par la présence de 2 équivalents temps plein sur toute la saison d'ouverture de l'Exposition de début mai à fin octobre malheureusement début août 2022. Météo France par l'intermédiaire du directeur de l'interrégion Sud-Est a fait part à la communauté de communes de la forte diminution du personnel, mise à disposition. À quelques mois de la libération prévue à mai 2023, après 5 années d'études et de travaux, le projet sera fortement remis en question. À compter du 31 août 2023 et les élus gardois témoin de cette situation ne savent plus à qui ils peuvent accorder leur confiance dans le contexte actuel d'urgence climatique de crise énergétique. Je ne comprends pas ce désengagement et vous demande de bien vouloir soutenir ce projet auprès des instances de météo France. Je vous remercie. La mise en place du Centre du Mont Aigoual résulte. D'un long partenariat entre la communauté de communes et météo France l'établissement continuent d'acier. À la fois hein maintenant des personnels sur le site jusqu'à l'ouverture du Centre d'interprétation du changement climatique, prévue au printemps 2023 et en mobilisant plusieurs de ses spécialistes du climat pour participer au comité scientifique chargé de valider les contenus de la future muséographie. Météo France a toutefois connu depuis 10 ans une réduction de ses effectifs de plus de 25% et une restructuration de ses implantations territoriales avec la fermeture de tous les centres départementaux. Météo France a donc été amenée à mettre fin à la mise à disposition d'effectifs permanent pour des missions d'animation scientifique dans tous les lieux où l'établissement était présent au niveau national, notamment à La Villette à Paris ou encore à la Cité de l'espace à Toulouse. malheureux n'est donc malheureusement plus en mesure de mettre du personnel à disposition pour l'animation scientifique du Centre du Mont Aigoual. Dans le cadre de son plafond d'emplois actuels, que ce soit contre remboursement par les collectivités Comme cela avait été envisagé, notamment en 2008 2019 ni gratuitement comme le demande la communauté de commune Causses Aigoual Cévennes pour aider au financement au lancement du Centre météo France propose toutefois d'apporter un appui au cours de la première saison l'ouverture dans le cadre d'un partenariat dont les modalités ont déjà fait l'objet de discussions localement. Compte tenu de l'importance de ce projet pour la communauté de communes et de l'engagement de météo France dans sa réalisation. La présidente directrice générale de météo France, devrait se rendre. Sur place prochainement pour venir échanger avec l'ensemble des élus concernés et acteurs de ce projet.-- Nous passons maintenant Madame Sollogoub qui a la parole. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre je souhaite vous alerter sur les difficultés que rencontrent les petites communes rurales, dans le cadre de leur participation aux dépenses communales de fonctionnement des écoles publiques accueillant des élèves dont la famille est domicilié dans une autre commune. L'article L 212 tiré 8 du code de l'éducation prévoit que lorsqu'une commune reçoit des élèves dont la famille est domicilié dans une autre commune. La répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence ce principe de libre. Accord dans la répartition des charges de fonctionnement entre communes d'accueil et commune de résidence connaît des réalités varier selon les territoires et les tarifs fixés se situe bien souvent au delà des possibilités financières des communes rurales les moins aisés. Le 3ème alinéa de ce même article prévoit certes la prise en compte des ressources de la commune de résidence dans le calcul de la contribution mais alors des réalités les communes d'accueil elles-mêmes ce sont parfois en difficulté pour faire face à leurs frais de fonctionnement qui sont de plus en plus élevé. Si bien que les les communes rurales. De résidence des enfants ce sont très souvent lésés. Alors je voudrais savoir si le gouvernement entend éventuellement aider les communes d'accueil dans leurs frais de fonctionnement ou fixer un barème de calcul qui tienne davantage compte des ressources réelles dont disposent les communes de résidence des élèves. Je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la ministre, votre réponse. Non. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les les sénateurs, madame la sénatrice ce logo. J'entends toute l'attention que vous portez aux contraintes financières des petites communes rurales ne disposant pas d'école et je la partage. Afin d'éviter certaines difficultés inhérentes aux communes rurales les moins peuplées, le code de l'éducation autorise 2 ou plusieurs communes à se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école et rend cette disposition obligatoire lorsque 2 ou plusieurs localités distantes de moins de 3 kilomètres la population scolaire de l'une d'elles est régulièrement inférieure à 15 élèves. Par ailleurs, le code de l'éducation mentionne que lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domicilié dans une autre commune. La répartition des dépenses de fonctionnement se fait par la par par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence et précise également que pour le calcul de la contribution de la commune de résidence. Il est tenu compte des ressources de cette commune du nombre d'élèves de cette commune scolarisé dans la commune d'accueil et d'une coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil les dépenses à prendre en compte à ce titre-sont les charges de fonctionnement à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Par voie de conséquence, les négociations relève des communes pour trouver un accord, tenant compte des éléments précisé dans cet article il n'entre pas dans les prérogatives du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse d'interférer dans ces négociations. Toutefois, à défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses. La contribution de chaque commune est fixé par le préfet après avis du conseil départemental de l'Éducation nationale. Ainsi ces dispositions permettent de répondre à l'ensemble des difficultés rencontrées et il n'apparaît donc pas opportun de mettre en place des aides compensatoires compensatoires compensatoires à destination des communes d'accueil en définitive je peux vous assurer que le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse attaché en matière d'école en milieu rural reste particulièrement vigilants aux dispositions qui régissent à la répartition et la contribution aux frais de fonctionnement des écoles notamment s'agissant des communes ne disposant pas d'école. Merci. Merci chère madame la ministre madame madame goût on peut continuer. Oui Madame la Ministre je voudrais quand même vous donner quelques exemples pour vous preniez la mesure du problème. Ah Amazit toute petite commune rurale de la Nièvre en 2010 il y avait 30 enfants, ils ont dû pas contribuer à hauteur de 30.000 euros aux frais de scolarité cette année la la commune n'a pas boucler son budget en 2022 à Manny l'orme pour 2 enfants en primaire et un en maternelle y contribue à hauteur de 4000 euros pour 2023 ans, leur annonce 10.600 euros pour 2024 16.700. Alors pour cette raison, il y a certaines communes rurales qui en sont à appréhender de voir venir des familles avec des enfants sur leur territoire ce qui je dois le dire dans un département déprise démographique démographique est vraiment un comble. Je vous remercie d'être vraiment attentive à ce sujet. Merci, merci, cher collègue, c'est un beau message pour le préfet de la Nièvre, me semble-t-il. Monsieur Pacaud à la parole.-- Merci monsieur le président, madame la ministre, hein. Je vais vous parler d'inclusion scolaire. Puis la loi de 2005 et même s'il reste encore beaucoup à faire d'énormes progrès ont été réalisés pour mieux accueillir au sein de l'école de la République des. Enfants frappés par le destin et par le handicap que s'en féliciter, mais surtout ne pas s'endormir sur sur nos lauriers pour faire mieux. Or, aujourd'hui, se pose un problème qui concerne désormais presque toutes les écoles de France, c'est l'accueil des élèves qui présentent des troubles du comportement et qui relèvent normalement de structures adaptée des IME ou des ITEP. Ou ses enfants bénéficient d'éducateur spécialisé. Or, les places dans ces structures s'avérant insuffisante l'éducation nationale a décidé depuis 2 3 ans, de les inclure au sein des classes traditionnelles ce qui s'avère catastrophique dans la plupart des cas avec notamment l'installation d'atmosphère délétère qui conduisent où peuvent conduire nombre de professeurs au bord de la dépression. Ou au bord de la démission. J'ai en tête bien des exemples de professeurs chevronnés, secondée par des AESH. Mais qui sont impuissants face à l'attitude agressive violente de certains de leurs élèves et qu'ils ne reçoivent aucune aide qui ne reçoivent aucune écoute de la part de leur hiérarchie. Ces situations sont aussi préjudiciable pour ses enfants en difficulté de comportement. Qui sont inclus là où il ne devrait pas l'être et qui s'y épanouissent rarement et elles sont aussi préjudiciables pour leurs petits camarades qui subissent ces conditions d'enseignement dégradés. J'ai alerté le ministre à plusieurs reprises, rien ne bouge. Ma question est simple, le gouvernement compte-t-il enfin cesser d'ignorer cette problématique et de donner à l'éducation spécialisée. Les moyens d'accueillir enfin tous ces enfants qui ne relèvent pas de structure traditionnelle. Merci cher collègue. Madame la Ministre votre réponse.-- Merci monsieur le le président, mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Paco le droit à l'éducation est un droit fondamental, c'est d'ailleurs pourquoi le président de la République a fait de la scolarisation des enfants en situation de handicap, une des priorités dès son premier quinquennat. Depuis 5 ans, des progrès sont notables et ils ont été obtenus aujourd'hui près de 476.000 élèves en situation de handicap sont scolarisés et 184.000 accompagnants ont été recrutés. Toutefois, en dépit de tous les ses efforts, nous devons encore progresser. C'est pourquoi en ce moment même les ministres. Pap Ndiaye et Geneviève Darrieussecq sont engagés avec tous les acteurs afin de définir un véritable acte de de l'école inclusive. Le président de la République annoncera au printemps des mesures ambitieuses particulièrement sur la question des élèves qui s'ouvrent de trouble du comportement. Après avoir échangé avec l'éthique, l'équipe éducative, la famille peut solliciter l'évaluation de la commission des des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en vue d'une reconnaissance de situation de handicap le cas échéant se voir attribuer des mesures de compensation les Ulis, constitue une des modalités de mise en oeuvre de l'accessibilité pédagogique, une carte des Ulis est arrêté annuellement par le recteur d'académie en concertation avec les directeur académique des services de l'éducation nationale, autrement appelé Dasen. L'objectif de cette carte et d'assurer un maillage territorial serré en cohérence et sa complémentarité avec l'offre médico-social et l'offre de soins pilotée par les agences régionales de santé depuis 2017, la politique d'ouverture de dispositifs Ulysse est une priorité du ministère grâce au volontarisme du gouvernement, nous en comptons désormais 10.300 et ancêtre entier. Rentrée 2022, nous avons ouvert plus de 300. Ulysse, les élèves présentant des difficultés à expression comportemental peuvent aussi être scolarisés en classe ordinaire et s'il bénéficie d'un projet personnalisé de scolarisation peuvent être accompagnés par un AESH vous l'avez précisé les dispositifs institut thérapeutique éducatif et pédagogique peuvent aussi répondre aux besoins de certains enfants, vous le voyez, nous avons à coeur de trouver une solution pour chaque élève, une solution qui soit la plus adaptée possible aux besoins de l'élève. Je vous remercie. Merci madame la ministre pour la précision et la brièveté de vos réponses. La parole est maintenant à monsieur Jean-Yves Roux.-- Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre. de réponse. Prend la parole pour trois secondes, mon cher collègue. Je vous remercie. Des annonces. J'ai noté qu'il y aurait une annonce présidentielle mais vraiment le trou du comportement n'est pas un handicap comme les autres, on manque 10 1000ème Edith. Merci président.-- Chers collègue Jean Véro.-- Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme beaucoup d'élus, nous sommes placés depuis quelques semaines face à la détresse de nos artisans de bouche, boulangers, bouchers, charcutiers, restaurateurs, traiteurs, confronté à la coalition d'une crise énergétique climatique et politique très inquiétante. Face à l'envolée des prix de l'énergie et des matières premières, ces artisans ne peuvent fermer leur four leur charme froide se passer de farines ou de beurre, pas plus commenté de mesurer ma leurs tarifs pour y répondre. Le gouvernement a proposé mardi dernier différentes mesures Alain de report d'imposition, la création d'un guichet unique ou renégociation de l'État avec les différents opérateurs en indiquant une aide pour le volet énergétique pouvant aller jusqu'à 40% des factures. Ces mesures sont bonnes à prendre. Pourtant chez nous un Alpes-de-Haute-Provence nos artisans, artisans boulangers un test nous disent d'ores et déjà que cela ne suffira pas à passer cette année et qu'ils ont besoin de plus de visibilité et de simplicité d'action. Et chers collègues et en particulier, mes chers collègues, de la ruralité nous savons plus que toute autre combien ces artisans de bouche sont essentiels à la vie de nos communes d'activités de proximité des boulangers, bouchers charcutiers traiteurs. C'est ce qui permet aussi à nos habitants, notamment les plus fragiles de ne pas faire des kilomètres pour s'approvisionner. C'est une garantie de manger des produits de qualité, c'est aussi l'assurance que la puissance publique considère équitable ma chacun de ces habitats hyper rural ou hyper citadelle. Monsieur le Ministre, tous les élus se battent chaque jour avec l'État, l'Europe pour soutenir et revitaliser nos petites communes et notre commerce de proximité. Or la disparition d'un artisan de bouche la ruralité peut sonner le glas d'années d'efforts conjoints une Messi se vend public, elle n'a pas la même signification. Monsieur le Ministre, seriez-vous prêt à proposer des tarifs réglementés plus avantageux à nos artisans notamment se présente dans les zones de revitalisation rurale le gouvernement est-il prêt à proposer des aides complémentaires au maintien des commerces ruraux au titre de la cohésion des territoires et ça à s'engager sur le moyen terme pour leur permettre d'investir durablement dans des modes de production moins énergivores et plus autonome. Je vous remercie.-- Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre.-- monsieur le président, Monsieur le Sénateur, je souhaite profiter de la question que vous m'adressez et des suivantes qui concerneront des sujets similaires pour refaire le point sur les aides mises en place pour nos entreprises face à la hausse du coût de l'énergie et notamment les plus petites d'entre elles plusieurs dispositifs sont mises en oeuvre, comme vous le savez, d'abord le bouclier tarifaire sur l'électricité TPE. Ont TPE de moins de 10 salariés et 2 millions de chiffre d'affaires ayant un compteur électrique d'une puissance inférieure à 36 kilovoltampères elles sont éligibles en 2022 et 2023 au bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité qui va donc s'établir à 15% en moyenne pour pour cette année. Les fournisseurs d'énergie sont par ailleurs engagés à fournir à leurs clients TPE non éligibles au bouclier tarifaire des contrats ou le coût de l'électricité ne dépasse pas les 280 euros. Du mégawattheure les modalités d'application de cet engagement sont en cours de précision. Troisièmement l'amortisseur électricité à partir de 2023 pour les les PME. Toutes les TPE qui ne sont pas protégés par le bouclier tarifaire et toutes les PME bénéficient d'un nouveau dispositif d'amortisseur électricité l'État prend en charge une partie de la facture ce montant est déduit afficher directement sur la facture de l'entreprise et puis enfin, l'aide au paiement des factures des très très cité et de et de gaz. À laquelle peuvent bénéficier les les entreprises. Jusqu'à 4 millions d'euros, c'était d'être accessible sur le site impôts Point pour le mois de septembre et octobre 2022, le guichet demandait d'être ouvert depuis le 19 novembre et pour les périodes suivantes, il sera ouvert le 7 janvier 2023. En 2023, cette aide peut être demandée par les TPE et PME qui ont bénéficié de l'amortisseur dès lors qu'elles ont respecte les critères les deux dispositifs permettront une prise en charge par l'État de 35 à 40% de la hausse de la facture. Cette mesure concerne précisément les publics que vous mentionnez dans votre question, la possibilité pour certaines entreprises dont les boulangers de demander le report du paiement des impôts et cotisations sociales. Comme annoncé par la Première ministre de la semaine dernière et la dernière des mesures que je voulais citer le temps qui m'est imparti ne permet pas de développer davantage mais je voudrais simplement. Rappeler que pour celles et ceux qui ne se retrouveraient dans aucun de ces dispositifs. Il leur appartient de se rapprocher du conseiller départemental. Sortie de crise qui pourra essayer d'apporter des solutions complémentaires.-- Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le mis c'est vous. tous les autres points au sur les quais sont arrivés les antennes des opérateurs télécoms. La multiplication de ces pylônes. Porte à l'évidence atteinte au paysage et provoque crainte et mécontentement de nombre de nos concitoyens. Ce mitage du territoire ne règlent d'ailleurs pas le problème persistant de zones blanches dans notre pays et notamment dans mon département de la Somme. Après plus de 20 ans de patience. On se demande d'ailleurs comment il est possible en 2023 que son portable puisse encore être coupé à tout moment dans un territoire alors même que paradoxalement nous battons les records d'installation téléphonique on peut échanger en Direct avec Thomas Pesquet basé à 400 kilomètres en orbite son arrestation ISS mais d'un village à l'autre ça bug. L'explication de cette situation ubuesque réside notamment dans notre incapacité à mutualiser ses installations et notamment les relais téléphoniques, selon l'Agence nationale des fréquences, plus de 300.000 antennes relais déjà notre territoire certes des partages d'infrastructures entre opérateurs existe déjà et fonctionne bien, cela permet aux opérateurs de partager à matériel existant et donc d'éviter des doublons d'infrastructures et d'assurer ainsi une couverture optimale du territoire. Monsieur le Ministre, afin de lutter contre les fractures territoriales. Le gouvernement prévoit-t-il des mesures plus incitatives et pourquoi pas et je pense que ce serait bien plus contraignante en faveur de la mutualisation des pylônes et des antennes relais par les opérateurs, ce serait à mon avis une étape essentielle pour lutter très efficacement contre les déserts téléphonique.-- Monsieur le Ministre, là vous êtes dans votre coeur de métier. Merci monsieur le président, monsieur le sénateur, et effectivement il y a là une forme de. D'injonctions Il s'agit à la fois de résorber les les zones blanches mais évidemment d'éviter la multiplication des antennes qui ont une une empreinte. Carbone qu'il convient de. le principal outil dont dont nous disposons pour inciter à la mutualisation, comme vous le savez c'est le New Deal mobile qui a été conçu il y a à peu près 5 ans. Pour effacer en à l'horizon 2027 5000 zones blanches dans notre pays en imposant ou en exigeant de la part des opérateurs, que sur les pylônes New Deal qui se serait attribué pendant cette période. Là les les pylônes cette les pylônes soient mutualisés et donc les 5000 antennes New deal qui vont se déployer jusqu'en 2027 sont effectivement. Mutualisées et ont permis pour les 2000. Qui sont d'ores et déjà installés d'effacer progressivement les zones blanches dans notre pays, d'autres obligations légales sont déjà en application, comme l'obligation en zone de montagne, ou dans le cadre du déploiement 5G en zone peu dense. Enfin la loi du sénateur Patrick Chaize visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique notamment son article 30 oblige les opérateurs à justifier auprès du maire, du choix de ne pas recourir à une solution de partage du site. Ou de pilotes grâce à l'ensemble de ces mesures. L'Arcep indique dans le cadre de son rapport annuel que 70% des antennes sont sont mutualisés. Nous continuons nos efforts pour garantir une couverture de l'ensemble de nos concitoyens. 600 sites New Deal vont être couvert pour l'année 2023 donc 600 sites mutualisés. Il en sera de même pour les 2 prochaines années pour votre département de la Somme, 30 sites ont été identifiés depuis le début du dispositif et 4 nouveaux sites sont attribués pour. 2023 des sites mutualiser donc les opérateurs de télécoms se sont en également engagé à une couverture des axes prioritaires et ferroviaire ainsi que d'assurer une couverture nécessaire à l'intérieur des bâtiments, des trains et dévoile voilà monsieur le sénateur. Quelques éléments de réponse à votre question.-- Merci beaucoup monsieur le Ministre, la parole est maintenant Monsieur Guillaume Chevrollier.-- Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, dans nos communes et les petits commerces de proximité sont inquiétés menacé par la crise énergétique. Confrontée à une hausse du montant de leur facture d'électricité avec des montants multiplié par quatre. Pas par 10 ces professionnels sont de plus en plus résigné et certains envisagent de cesser leur activité. Un exemple dans mon département de la Mayenne avec une boulangerie qui n'a d'autre choix que de mettre la clé sous la porte, notamment en raison d'une facture d'électricité qui passera de 11.000 euros en 2022 à 41.000 euros en 2023. C'est le cas des des boulangeries de tous les métiers de bouche, mais aussi des des garagistes pour soutenir ces commerçants artisans. L'État a fait de nombreuses annonces et mis en place de nombreuses. La dernière en date étant le plafonnement à 280 euros du MWh pour les les TPE, ce qu'il y a encore beaucoup pour certains, mais ce que les entrepreneurs demande aujourd'hui, c'est de la visibilité. Depuis plusieurs mois avec d'autres collègues on a relayé auprès du gouvernement. L'inquiétude face à des mesures qui n'étaient pas adapté le temps leur a donné raison. Est ce que des ajustements dernières minutes. Ont été faits, ils font planer un climat un peu de de confusion. De plus, la profusion d'annonces contribue à renforcer ce manque de de compréhension par les professionnels qui se retrouvent à à devoir naviguer au milieu de démarches administratives complexes complexe chronophage et qui évolue presque du d'une semaine à à l'autre. Alors nos artisans commerçants et souhaite. Aussi une visibilité sur l'action du gouvernement dans la durée. Au regard de toutes les aides disponible et auquel elles ont accès les TPE doivent pouvoir juger de leurs perspectives d'avenir si elles peuvent continuer leur activité si elle doit se réorganiser embauché ou pas des apprentis. Et enfin, puisque cette qui semble s'installer dans la durée, ne faut-il pas également s'interroger sur la nécessité d'orienter les aides vers l'achat d'équipements moins énergivores, plutôt que de distribuer des aides à fonds perdus. Je souhaiterais donc savoir quelles actions le gouvernement compte-t-il prendre, afin de garantir cette visibilité et et cette clarté à tous nos commerçants artisans qui sont au coeur du lien social dans le territoire particulièrement dans les territoires ruraux. Nous devons les protéger et en rappelant que ces entrepreneurs ne veulent pas vivre de subventions, mais des fruits de leur travail. Je vous remercie. Si cher collègue, Monsieur le Ministre. Merci monsieur le le président, monsieur le sénateur, pour apporter de manière pérenne une une visibilité à aux entreprises de France s'agissant du prix de l'énergie. La stratégie qui est celle du gouvernement c'est d'une part. délais de d'énergies. Décarbonnées française. C'est tout l'objet du projet de loi sur les énergies renouvelables. Qui a été discuté récemment. C'est tout l'objet du programme. Que nous entendons mener sur la filière nucléaire et puis, en parallèle de réformer le marché européen de l'énergie pour découpler le prix du gaz et de l'électricité et ramener le prix de l'énergie à un niveau qui est plus proche de son coup en tout cas. Du coup, telle qu'il telle Dans sa fabrication en France. Ceci étant dit, il y a des des sites. Situation telle que celle que vous évoquez qui appelle à un accompagnement tout particulier et sans revenir sur les les mesures qui ont été évoqués simplement rappeler que le ministre de l'Économie et des Finances. La ministre déléguée en charge des PME du commerce et de l'artisanat ont réuni à plusieurs reprises des organisations représentatives des boulangers, notamment le 25 novembre et et le 3 janvier dernier, mais plus généralement les fédérations professionnelles Notamment mis un, un certain nombre de dispositifs en place pour. Apporter une une réponse au plus près du des des entrepreneurs de France, le médiateur de l'énergie peut accompagner les TPE dans leurs échanges avec les fournisseurs d'énergie, notamment en cas d'inquiétude sur des clauses contractuelles. Le médiateur des entreprises est quant à lui le point de contact des PME dans. Dans leurs relations avec les fournisseurs d'énergie le conseiller départemental à la sortie de crise accompagne les les entreprises dans la mise en oeuvre de de ces aides et et je précise que le numéro de portable des conseillers départementaux à la sortie de crise est disponible sur le site internet, ministère de l'Économie et des Finances et enfin les consulaires et ont été mis à contribution les CCI vont appeler appeler au téléphone 20.000 entreprises en France et les CM1 vont appeler l'ensemble des 33.000 boulangeries de notre pays pour leur faire connaître tous les dispositifs à leur disposition. Merci, monsieur le Ministre, la parole est maintenant à monsieur Christian Klinger. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, de la souveraineté industrielle et numérique au sujet de l'automatisation. Du fonds de compensation de la TVA. Certaines dépenses sont devenus inéligible pour les collectivités. C'est une perte sèche qui déséquilibre financièrement les projets concernés. Cette perte du FCTVA pour l'ensemble des dépenses d'acquisition et d'aménagement de terrain par exemple, va à l'encontre du soutien à l'investissement local d'autant plus important dans un contexte de relance de l'économie. À titre d'exemple pour la ville de Münster le programme d'investissements pour 2022 comportait. Un important projet d'aménagement de terrain de football pour un montant de 770.000 euros. Ce projet offrira au club de football local là est master des conditions d'entraînement amélioré mais également à tous les scolaires de disposer d'un équipement moderne pour l'enseignement sportif. Dans le dispositif de FCTVA avant automatisation cet investissement aurait été éligibles au FCTVA et t'aurais et aurait ainsi généré une recette d'investissement de 126.300 euros en année N plus Aujourd'hui ce manque à gagner, du fait de la réforme du FCTVA est préjudiciable pour les finances communales et pour le contribuable puisque c'est de l'emprunt qui devra s'y substituer. Pour financer cet important projet d'investissement sportif. Les communes ont donc un manque à gagner important qui ne leur permet plus d'équilibrer les opérations lancées. Ma question est très simple. Comptez-vous procéder à la réintroduction d'urgence des opérations d'aménagement et d'acquisition de terrains dans le Champ du FCTVA réintroduction qui avait été voté par le Sénat lors de l'examen du PLF 2023.-- Pense du gouvernement, Monsieur le Ministre.-- Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur, la loi de finances pour 2021, mettent en oeuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée le FCTVA pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure manuelle, dans le cadre de laquelle les collectivités devait déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution du FCTVA par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA. s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soient préservés pour autant le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire des ajustements ont dû être opérée dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Le compte 212 agencement et aménagement de terrain n'a pas été retenue dans l'assiette des car il ne comporte des dépenses hors taxes. Qui sont nécessairement inéligible au FCTVA par ailleurs le compte. 2051 concessions et droits similaires brevets licences Marc procédé logiciel droits et valeurs similaires ne fait pas non plus partie de la nouvelle assiette automatisé car il enregistre des dépenses inéligibles. Oui c'était bien. À sujet il convient de noter que le gouvernement a élargi l'assiette du FCTVA aux dépenses de service de l'informatique en nuage selon un taux de 5,6%, par amendement à la loi de finances rectificative pour 2020. Depuis le 1er janvier 2021. En août, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités notamment en supprimant le non recours ou FCTVA pour plusieurs dans d'entrée lors de sa première année de mise en oeuvre cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires en prenant en compte la prévision du FCTVA 2022 à 6, 5 milliards d'euros. 69% a été versé au 1er septembre, soit près de 4,5 milliards. L'année dernière à la même date, seulement 42% du total de l'attribution 2021 avait été décaissés considérée dans sa globalité la réforme de l'automatisation s'avère donc favorable à l'investissement public local. Toutefois, dans le cadre des débats parlementaires du projet de loi de finances pour 2023, le ministre délégué aux comptes publics a indiqué qu'un bilan de la réforme de l'automatisation du FCV TVA sera conduite. Une fois que la dernière partie des collectivités aura basculé dans l'automatisation, soit dans le courant de l'année 2023.--

Monsieur le Ministre, je regrette tout de même fortement que la réintégration de ces opérations. N'ait pas été. Concluante hein lors du du PLF d'autant plus que le ministre en séance avait laissé entendre qu'un accord pouvait être possible sur ce point. C'est une mesure qui est très attendu par par les maires. J'ose espérer que vous allez changer de position

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur l'impact de l'envolée des coûts de l'énergie pour les entreprises, en particulier pour les plus petites d'entre elles, et notamment les boulangers. Malgré les dispositifs d'aide mis en place ces professionnels subissent durement les conséquences de la crise énergétique qui s'ajoute aux augmentations conséquentes des tarifs de matières premières. Confronté à des prix de l'électricité et du gaz qui explose les entreprises grandes consommatrices d'énergie ou celles qui doivent renégocier leur contrat souffre et beaucoup voient leurs équilibres économiques menacés en France les entreprises mais je pourrais également y associer les collectivités bénéficiant d'un abonnement électrique supérieure à 36 qui avait ah ne peuvent pas accéder ou revenir au tarif réglementé de vente d'électricité plus protecteur et constituant un excellent bouclier tarifaire. Ce plafond 36 avait a prévu dans la loi française exclut de facto une part significative des quelque 30.000 boulangers et plus largement tous les sites de consommation raccorder sous une puissance souscrite supérieure à ce seuil. Ce critère de puissance et en aucun cas imposée par le droit de l'Union européenne et la France pourrait donc décider librement de le supprimer. C'est pourquoi je souhaite savoir si le gouvernement envisage d'agir en ce sens afin de permettre aux consommateurs professionnels d'électricité de petite taille de bénéficier également des tarifs des tarifs réglementés pour leur site raccordés sous une puissance souscrite à 36 Kader. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre.-- Merci monsieur le président, monsieur le sénateur, comme vous le savez et comme vous l'avez rappelé les les TPE dont la, la puissance installée. Est inférieur à 36 kilovoltampères bénéficient de ce bouclier tarifaire qui limite la hausse des prix pour 2023 à 15% après l'avoir limité à 4% pour l'année 2022 qui ne sont pas éligible à ce bouclier pour la puissance installée supérieure à 36 kilovoltampères. Elle bénéficie du dispositif d'amortisseurs ce dispositif d'amortisseur de toute évidence n'était pas suffisant et c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, le gouvernement a. Annoncé que toutes les TPE qui ont un contrat signé au 2ème semestres 2022 dont le prix moyen annuel de la part énergie pour 2023 dépasse 280 euros du MWh verront leur prix, le prix de leur contrat plafonné à ce niveau-là. En 2023, les TPE devront se signaler auprès de leur fournisseur d'électricité pour bénéficier de ce dispositif en remplissant l'attestation disponible sur le site impôts Point gouv Point FR ou auprès du fournisseur d'électricité. Par ailleurs, depuis le 1er janvier, juillet 2022, une aide d'urgence gaz électricité a été mise en place le dispositif a été prolongé jusqu'à fin 2023, il a été simplifiée notamment pour les aides de faible montant, c'est-à-dire les aides allant jusqu'à 4 millions d'euros. Vous savez qu'il y a un palier à et un autre à 150 millions d'euros pour en bénéficier de critères doivent être satisfaits. Les dépenses d'énergie de l'entreprise atteignent 3% de leur chiffre d'affaires de 2021 et le prix unitaire moyen du mégawattheure payé par ces entreprises a augmenté d'au moins 50% par rapport à l'année 2021. En parallèle, comme je le disais en introduction, toutes les TPE qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire et les PME sont éligibles. Depuis le 1er janvier 2023 l'amortisseur électricité cet amortisseur prend en charge 50% de la part énergie de la facture dans une fourchette de prix de 180 euros à 500 euros du MWh pour bénéficier de l'amortisseur électricité les entreprises doivent impérativement se déclarer éligible auprès de leurs fournisseurs et c'est au niveau de leur facture que se fait la déduction si je puis dire. Par ailleurs, je veux rappeler que. À disposition de toutes les entreprises se trouvent les conseillers départementaux à la sortie de crise dont les numéros de portable, les numéros de fixes sont désormais affichés sur le site internet du ministère. De l'économie De l'économie et je veux vous assurer en conclusion, monsieur le sénateur, de pleine mobilisation pour préserver notre tissu économique dans cette période. Les règles actuelles les règles qui ont été mis en oeuvre. Néanmoins ma question portait sur le pourquoi on n'arrive pas à faire en sorte de déplafonner ce 36 qui avait à et de faire en sorte que le bouclier tarifaire puisse s'appliquer sur l'ensemble des tarifs. Qui donc sont aujourd'hui il est plus fréquent dans les entreprises. L'amortisseur. Évidemment c'est toujours mieux que rien mais n'est pas suffisant de façon très claire aujourd'hui vraiment on a des des des des artisans qui qui. Mettent la clé sous la porte parce qu'ils ne peuvent pas. et je pense que très franchement j'entends que la mesure a un coût mais que ce coup il faudrait le mesurer le comparer au coût que coûteront. Ben les problématiques de toutes ces entreprises qui ne pourront plus produire et qui du coup n'apporteront pas leur. leur fiscalité dans dans le budget de de l'État. Donc je vous invite vraiment Monsieur le Ministre, à voir ce point là parce que ça serait vraiment une solution qui serait appréciée. Merci, cher collègue, la parole maintenant à Madame Darcos. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, l'actualisation des paramètres d'évaluation des valeurs locatives de des locaux professionnels qui sert d'assiette pour l'établissement des impôts Directs locaux a suscité l'année dernière la vive inquiétude des élus et des chefs d'entreprise dans mon département, l'Essonne et commissions intercommunales des impôts Directs. C'était très vite trouvé dans l'impossibilité de prendre un avis éclairé dans le délai de deux mois qu'il aurait été légalement impartis. De nombreux maires nous avait même par ailleurs signalé la probabilité de forte augmentation de la fiscalité locale. Ces augmentations étaient d'autant moins compréhensible qu'elle concernait en 1er lieu les commerces de centre-ville ou de centre-, bourg que nos municipalités s'efforce de préserver coûte que coûte. La loi de finances pour 2023 a tiré les leçons des difficultés rencontrées par les commissions locales pour mener à bien leurs travaux et a prévu le report à 2025 de l'entrée en vigueur des nouvelles bases d'imposition aussi des impôts locaux payés par les entreprises. Indéniablement sur ce report est né c'est au regard du caractère extrêmement parcellaire des données utilisées pour l'actualisation des paramètres collectif d'évaluation et du besoin pour les commissions départementales des valeurs locatives d'une plus forte visibilité sur les conséquences de leur décision. Il s'agit à présent de définir les modalités selon lesquelles les travaux d'actualisation pourront être poursuivis dans la perspective de leur intégration au bases d'imposition pour l'année 2 sont 2025 ans toutes cause il sera nécessaire d'associer étroitement les élus locaux et les entreprises contribuables dans le cas de cette démarche. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre m'apporter toutes les précisions utiles sur le calendrier et la méthodologie envisagez vous comprendrez parfaitement que nous devons aux élus et aux entreprises de nos territoires. La plus grande transparence et l'information la plus exacte possible. C'est la condition sine qua none du consentement à l'impôt. C'est pour ça que ma question n'est pas obsolète par rapport aux annonces de de de le dernier projet de loi de finances, je vous remercie de votre réponse. sur ce sujet important non seulement pour les finances des collectivités mais aussi, et vous l'avez rappelé, pour les entreprises la sont nationale et le sénat ont en effet décidé en loi de finances pour 2023, d'un report de 2 ans de l'actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Je tiens à rappeler que ces valeurs locatives ont été révisés en 2017 dans l'objectif que les impôts foncier soit établie au plus près du marché locatif. Il s'agit d'un succès important et l'actualisation régulière de ses bases révisé et l'un des éléments fondamentaux qui pourront garantir que les impôts fonciers sont répartis équitablement entre les entreprises, comme vous le rappeler, la révision de 2017 a été accompagné par plusieurs mécanismes destinés à en juguler les effets. Tout d'abord le dispositif dit de neutralisation a assuré que la révision s'effectue à niveau de recettes constant pour chaque communes et EPCI et chaque impôt. Il a ainsi assuré que la révision ne se traduise pas par une augmentation généralisée de la pression fiscale sur les entreprises. Ensuite, pour lisser les évolutions avis individuelle l'augmentation brute des bases a été réduite par l'application d'un mécanisme appelé plan chaudement applicable jusqu'en 2025, tandis que l'augmentation d'impôts elles-mêmes a été lycée pendant une période de 10 ans, l'ensemble des ces mécanismes compte tenu de leur incidence sur le montant de l'impôt relève de la loi c'est pourquoi compte tenu de la décision du gouvernement de reporter l'entrée en vigueur de cette actualisation de tels mécanismes n'ont pas été à nouveau proposé au législateur sur ce point je tiens à rappeler que le choix qu'a fait le gouvernement découlent notamment des alertes émises par nombre d'élus sur les conséquences potentiellement importante de cette actualisation dans une période de fortes tensions économiques ainsi que sur le manque de visibilité laissée aux commissions locales des impôts chargée de se prononcer sur les nouvelles valeurs locatives les craintes que vous exprimez ont donc été madame la sénatrice, au vu de cette expérience. Le gouvernement a annoncé, lors des débats sur le de finances 2023 que toute avancée sur ce sujet devrait prendre la forme d'une concertation approfondie, au cours de l'année 2023 avec les entreprises et avec les collectivités qui partage l'objectif d'une meilleure répartition des impôts fonciers. Je vous remercie.-- Il vous reste quelques secondes, madame Barco si vous voulez. Non non mais. Merci monsieur le ministre est en effet on sera très vigilants. Vous comprenez bien que les DGFIP. Dans nos départements ont besoin aussi d'avoir un calendrier pour pas qu'on soit de nouveau au pied du mur. Comme la dernière fois et et être bousculée à devoir faire ses réunions auxquelles j'ai assisté. En 2 mois 3 mois où c'était un peu la panique. Madame Estrosi Sassone. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre, ma question porte sur la lutte contre la fraude dans le secteur de la rénovation énergétique. Si des mesures ont été mises en place avec l'ajustement du Label reconnu garant de l'environnement RGE. L'encadrement des certificats d'économie d'énergie, les échanges d'informations entre les administrations commune police Urssaf Tracfin Anna l'interdiction du démarchage téléphonique ou ou la mise en place de la plateforme en ligne Signal conso pour dénoncer des pratiques douteuses. Force est de constater malheureusement que des abus persistent, selon la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes qui contrôle les pratiques commerciales et les enquêteurs de police les fraudes à la rénovation énergétique représente une délinquance de proximité ciblant le plus souvent des personnes âgées ou fragiles, cette criminalité s'organise, notamment par l'achat de fichier clients à des centres d'appels puis au travers d'entreprises généralement titulaires de la mention RGE qui sous-traitent et qui pour certaines d'entre elles ne fonctionne que par le biais de boîte postale difficiles à identifier et à sanctionner en outre la fraude touche également les ménages qui pensent faire appel à des entreprises de bonne foi, comme en témoigne une enquête récente qui met en lumière un taux de non-conformité travaux qui atteint 51% pour les isolation des combles et 30% pour les isolation murale. Alors Monsieur le Ministre, quel est le bilan de la lutte contre la fraude au ces 2 E qui est au coeur des dispositions de la loi climat et résilience, comment entendez-vous améliorer la qualité des travaux et prévoyez-vous d'élargir la palette des contrôles. Enfin, les sanctions administratives et pénales et la collaboration qu'elles impliquent entre l'autorité administrative ou judiciaire. L'Ademe Elana sont-elles véritablement effective et efficace. Chers collègues. Merci Monsieur le Ministre pour cette réponse. Merci monsieur le président, madame la sénatrice. Le gouvernement et particulièrement attentifs à la protection économique du consommateur dans le secteur de la rénovation énergétique, notamment s'agissant des travaux de rénovation initiée par nos concitoyens, afin de limiter leurs dépenses d'énergies. C'est pourquoi nous avons mobilisé la DGCCRF sur cette problématique pour l'année 2023 un programme de contrôles renforcés ciblés prévoyant 1200 contrôles d'établissement est prévu. Je peux vous assurer que les suites appropriées seront données aux anomalies aux manquements relevés et que des suites pénales seront données lorsque des pratiques trompeuses seront mises en évidence ces contrôles portent déjà leurs fruits. À titre d'exemple, à la suite d'une enquête de la DGCCRF. Le gérant d'une entreprise a été condamné en décembre dernier pour pratique commerciale trompeuse à 12 mois de prison avec sursis probatoire pendant 3 ans par le tribunal judiciaire de Strasbourg. Il lui a en outre été interdit de gérer une entreprise pendant cinq ans et il devra verser aux parties civiles. Plus de 60 mais 67.000 euros de préjudice matériel et moral ainsi qu'on frais de justice. Par ailleurs, en s'appuyant sur les possibilités offertes par la loi climat et résilience, les services de l'État ont renforcé leurs échanges d'informations pour accroître la réactivité et l'efficacité de la lutte contre les fraudes. C'est le cas en particulier de la DGCCRF de Lana de l'Ademe et du pôle national des certificats d'économie d'énergie au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui sont très actifs dans ce domaine. Les services de l'État communique également aux organismes délivrant une certification une qualification. Les éléments recueillis à l'occasion de leur contrôle les entreprises aux pratiques déloyales ou frauduleuses peuvent ainsi se voir retirer le Label RGE de manière plus rapide. Enfin sur le sujet du démarchage téléphonique qui constitue un point d'entrée privilégié des acteurs les moins scrupuleux. La loi du 24 juillet 2020 a posé le principe de son interdiction totale dans le secteur de la rénovation énergétique, sauf en cas de contrats en cours. La DGCCRF a déployé un plan de contrôle spécifiquement axée sur le respect de cette disposition législative et plusieurs sanctions d'un montant dissuasif dépassant dans certains cas les 100.000 euros. À ce titre, ont d'ores et déjà été prises pour veiller à faire respecter ces dispositions. Puis donc vous assurer que les services de l'État sont pleinement mobilisées, c'est indispensable. Vous l'avez rappelé, pour protéger les consommateurs, pour garantir aux aux nombreux artisans honnêtes et compétents du secteur une concurrence loyale et pour permettre à notre pays d'atteindre ses objectifs climatiques ambitieux. Monsieur le Ministre Mesdames Estrosi Sassone. Merci Monsieur le Ministre, c'est indispensable également pour pouvoir véritablement passer à une massification de la rénovation énergétique. Donc je vois que le gouvernement est mobilisé, mais si j'ose dire, il ne faut absolument rien lâcher parce qu'il en dépend aussi des objectifs que nous pourrons toutes et tous se tenir pour nos concitoyens et pour permettre cette rénovation énergétique est absolument indispensable dans notre pays. Merci cher collègue. Je vais suspendre la séance sera reprise à 14h 30 pour l'examen de la proposition de résolution à l'application de l'article 34 1 de la Constitution proposant gouvernement de sortir le système électrique des mécanismes concurrentiels. Rien que ça. La séance est un suspendu.